La séance est reprise, nous reprenons la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après un engagement de la procédure accélérée pour un État au service d'une société de confiance dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 3 bis à à. à cet article, nous avons un 1er amendement numéro 38 qui est présenté par Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, il s'agit d'un amendement de suppression et ce pour 2 raisons : d'abord pour rappeler que les mesures fiscales ont leur place en loi de finances, inondant les lois ordinaires, de manière à favoriser une certaine cohérence de la politique fiscale et ainsi, l'article 3 bis à telle que rédigée ne relève à sous nos yeux, manifestement pas du Champ de la loi que nous examinons aujourd'hui sur le fond. Cet article additionnel a pour objet de préciser que le taux réduit de TVA, de 10 pourcent sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien est applicable dès le 1er raconte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de TVA soit fournis lors de la facturation finale au-delà Chevement des travaux, cette disposition est satisfaite par ailleurs puisque la doctrine puisque fiscal pardon prévoit déjà afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles en professionnels et particuliers qui fait réaliser des travaux de ne pas alourdir les charges administratives pesant sur les entreprises, que le taux réduit TVA s'applique dès le 1er raconte, sous réserve que les travaux et locaux soient éligibles dans la mesure où la disposition visé par cet article additionnel satisfaite et au auparavant hier, nous considérons que les mesures fiscales doivent trouver leur place en loi de finances et non pas en parloir, c'est une demande de suppression de cet article. Merci monsieur le ministre, avis de la commission Madame Bruni-. Merci madame la présidente. Je voudrais dire tout de soude bord que si vous dites que c'est cette amendement devrait être dans la loi de finances, je pense qu'il y a la moitié des articles en fait qu'on pourrait enlever, c'est un vrai droit à l'erreur ici, dont on parle. Donc cet article adopté par la commission spéciale visant à inscrire dans la loi une souplesse qui est déjà admise par la doctrine, c'est une mesure de sécurité juridique, il n'y a absolument pas lieu de s'y opposer pour mémoire pour bénéficier du taux de TVA réduit sur les travaux d'amélioration des locaux d'habitation, le client doit remettre à l'entreprise avant le début des travaux, une attestation mentionne à mentionnant que ces locaux sont achevés depuis plus de 2 ans, il est vrai qu'en pratique, l'attestation et parfois remise après le début des travaux ou le versement des premiers acomptes, ceci dit, la doctrine prévoit déjà une tolérance à ce sujet, elle dit, afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre les professionnels et le particulier et de ne pas accentuer la charge administrative pesant sur les entreprises, il est admis que le taux réduit de TVA s'applique dès le 1er raconte, sous réserve que l'attestation soit fournis lors de la facturation finale ou de l'achèvement des travaux, l'article 3 bis à vise à inscrire cette forme de droit à l'erreur directement dans la loi, cet article est issu d'un amendement de mon collègue Philippe. Sous-amendé par moi-même, donc avis défavorable pour la suppression de cet article. Merci madame la rapporteure je mets donc on voit l'amendement 38 E présenté par le gouvernement qui a donc un avis défavorable de la commune. Sion, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient l'amendement 38 n'est pas adopté, je mets donc on voit l'article 3 bis à qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, l'article 3 bis a est adoptée, je mets au voile, article 3 bis à qui est pour. C'est con. Qui s'abstient, l'article 3 bis a est adoptée article 3 bis. Nous avons un amendement numéro 133 qui est présenté par Monsieur merci madame la présidente, très brièvement, c'est un article suppression un amendement de suppression de l'article 3 bis article qui met en question quand même l'un des éléments essentiels de la lutte contre la fraude et la délinquance financière, puisque ça concerne le régime des provisions comptables qui parfois constitue un gisement important de dissimulation de certains résultats donc la confiance n'excluant pas la vigilance, nous proposons de supprimer cet article. Merci, cher collègue, avis de la commission c'est Madame Bruni qui rend la vie. Merci madame la présidente, les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés doivent transmettre à l'administration fiscale, une série de documents justificatifs suivi des rectifications dans les groupes intégrés, suivi des des plus-values latentes Tableau des des provisions, etc, en cas de défaut de transmission dans les délais ou d'inexactitudes une amende fiscale égale à 5 pourcent des sommes omise est appliquée toutefois la doctrine permet de ne pas appliquer cette amende si l'entreprise complète la transmission des documents, à condition que la démarche soit entièrement spontané, l'article 3 bis, adoptée à l'initiative de notre collègue député Véronique Louwagie vise à consacrer cette possibilité au niveau législatif et à l'étendre aux régularisations à la première demande de l'administration, il s'agit d'une mesure de bon sens qui encouragera la confiance mutuelle entre les entreprises et l'administration en fait ces ces documents ce ceux qui sont plutôt des des tableaux sont des annexes à ce qu'on appelle la liasse fiscale donc au au bilan et aux comptes de résultats et qui apportent en fait un complément d'information s'agit pas du tout du tout de documents qui permettent de calculer l'impôt, c'est juste un complément d'un information donc c'est pour ça que là c'est un vrai droit à l'erreur une omission et si est elle est comment revue spontanément et on vous demande de ne pas appliquer ces pénalités. Merci, avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, c'est le même avis que la Commission un avis défavorable, considérant que c'est un article qui a été introduit à l'Assemblée va dans le bon sens et permet d'établir ce lien de confiance donc, pour les mêmes arguments que ceux évoqués par Madame la rapporteur, l'avis est défavorable à la suppression. Très bien, merci Monsieur le Ministre, je mets donc voilà l'amendement 133 qui a un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est con. Qui s'abstient l'amendement 133 n'est pas adopté, nous passons à l'amendement 164 qui est présenté par Monsieur Philippe Dominati. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, dans le but de revenir à une relation de confiance entre les contribuables et l'administration fiscale, l'Assemblée nationale a tenté d'amender ce texte en introduisant l'article 3 bis puisqu'il estimait que le texte du gouvernement n'était pas suffisant le présent amendement a pour but de faciliter, d'une part, le travail de l'administration, en supprimant les certaines sanctions non modulable puisqu'il y a des sanctions ou des amendes disproportionnées par rapport à la faute, notamment lorsque par exemple la taxe ne bouge pas et que, en réalité, la base imposable ne bouge pas et que la sanction ou la taxe est égal à 0 0 euros mais vous payez l'amende, vous avez fait une faute, l'administration ne peut pas moduler la demande et si la base ne bouge pas, vous devez 0 au Fisc n'est pas comme vous devez l'amende alors le c'est en partie le but de cet amendement, ça se produit lorsque les bases sont égales à 0 ou ça se produit lorsqu'il y a une opération qui vient postérieurement à un an ou 2 ans après la déclaration, mais que ça ne change pas le but, encore une fois, de la somme que le contribuable doit payer au Fisc et lorsque le contribuable doit payer 0 au Fisc, mais qu'il doit payer une amende parce qu'il a manqué un papier parce que il a eu lieu, il n'était pas dans les délais, etc, l'administration elle-même n'a pas la possibilité de moduler cette amende, c'était le but de cet amendement, madame la présidente. Merci, cher collègue, avis de la commission. Madame Grenier. Merci madame la présidente, votre amendement ici sensiblement plus loin que la souplesse qui est admise par la doctrine et que l'article 3 10 prévoit de consacrer dans la loi, il s'agit de modifications très technique, hein, qui pourrait peut-être justifier sur le principe, mais dont les conséquences exactes sont difficiles à évaluer, alors on on propose en fait un retrait votre amendement, mais on aimerait bien entendre l'analyse du du gouvernement sur cette disposition aujourd'hui. Merci monsieur le ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présidente, l'amende prévue par l'article 1763 que vous évoquez, permet d'assurer le respect de l'obligation faite aux entreprises d'établir certains documents, notamment le registre suivi des plus-values, bénéficiant d'un report d'imposition, ce qui peut-être particulièrement intéressant à suivre, notamment dans le cas des restructurations de grandes entreprises, il s'agit de régimes fiscaux favorables dérogatoire au droit commun et dans les enjeux fiscaux peuvent être très élevés dans les cas que que j'ai votre rapidement, il faut donc préservé pour nous, la capacité de l'administration à suivre et contrôler ces dispositifs et nous considérons que l'assouplissement apporté adopté par l'Assemblée nationale est suffisant, qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin, comme vous le souhaitez, comme vous le proposez donc pour ces raisons, l'avis est défavorable, nous souhaitons rester à assouplissement apporté par l'Assemblée nationale.

nous passons à l'amendement 39 présenté par le gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, madame la présidente, il s'agit simplement d'une levée gages sur l'article.

Qui est. Qui s'abstient, l'article 3 bis est adopté article IV. Nous avons une demande de paroles de Madame Hélène Conway Mouret. Chers collègues, à vous la parole. Oui merci madame la présidente, madame et monsieur le rapporteur, mais monsieur le ministre, déjà, moi je voulais simplement exprimé une une grande déception de la part de mes collègues, cosignataire d'un certain nombre d'amendements que nous avons présenté qui se sont vus tous s'opposer l'article 41 alors que nous pensions nous inscrire complètement dans l'esprit de ce projet de loi pour faciliter les démarches administratives des usagers aussi faire gagner du temps, à la fois aux usagers, mais également à l'administration en pouvant hé bien avoir une bonne information mais surtout signalé aux 3 millions de Français que réside à l'étranger, et bien que l'État français ne les oublie pas et que la confiance est bien aussi doit régner avec ceux qui ont décidé de s'inscrire dans une mobilité avec 300000 Français qui partent chaque année 200000 qui rentrent en France et qui garde dernier un très fort avec ce pays, avec notre pays et qui ont besoin, hé bien, plutôt que de s'épuiser dans des démarches administratives souvent inutiles parce que il ne ne frappe pas au au bon guichet et multiplie les démarches hé bien pouvoir passer leur temps à trouver du travail et se réinsérer inscrire leurs enfants dans des écoles ce que nous avons essayé de faire par ces articles, et bien c'est de dire que voilà, nous pouvons aussi faciliter la vie de ceux la langue pour l'article 4 je voulais présenter un amendement dont l'intention était temps la procédure d'information de rescrit tout simplement auprès de l'administration fiscale prévues aux articles L. 80 elle 88 du livre des procédures fiscales, simplement parce que beaucoup de nos compatriotes qui partent à l'étranger et bien estiment à tort que leur situation fiscale est identique alors retour à celle qui était qui existait au moment de de leur départ et hé bien cette démarche leur permettrait de connaître les démarches éventuelles à effectuer pour se mettre en règle auprès de l'administration fiscale au moment de l'Europe, retour en France, je vous remercie. Merci, cher collègue. Nous passons à la présentation de l'amendement 134 ce monsieur, à madame pruneaux qu'il présente. Merci madame la présidente, chers collègues, nous proposons de supprimer cet article, en effet, nous considérons cet article comme la simple reformulation de l'article 62 duel PF alinéa 1 à 7, ajoutant en fait littéralement le cas des examens de situation fiscale personnelle à la liste des contentieux autorisant la régularisation spontanée un ajout au demeurant peu dispensateur de plus-values légal puisque l'article vise déjà l'ensemble des impôts de manière générique pour mémoire, la procédure ne concerne que 4000 contribuables par an qui dispose par ailleurs bien souvent de conseil juridique pour pour information, en 2016 les procédures concernées ont produit en moyenne plus de 175000 euros de rappel d'impôts à payer et 80000 euros de pénalités appliquées par comparaison les contrôles sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu, ont dégagé, pour leur part une moyenne de 3400 euros de droits, le reste de l'article n'apporte rien de plus au cadre existant, les articles L 80 et 80 B. duel PF définissant le rescrit fiscal et leur plus récente rédaction découle de la loi de finances rectificative pour 2017 promulguée en décembre dernier, je vous remercie. Merci, cher collègue à l'avis de la commission. Merci madame la présidente, ce sera un avis défavorable, l'article 4 contient plusieurs dépôts principales dispositions fiscales du texte, la réduction de 30 pourcent de l'intérêt de retard en cas de régularisation par le contribuable au cours d'un contrôle fiscal pour l'ensemble des procédures de contrôle, l'inscription dans la loi de la procédure de rescrit fiscal en cours de contrôle et surtout la garantie fiscale introduite par les députés et préservé par notre commission spéciale en vertu de laquelle tous les points examinés lors d'un contrôle et n'ayant pas fait l'objet de rose de réhaussement seront considérés comme tacitement validé par l'administration, tient absolument en fait à cet article donc avis défavorable. Si Madame la rapporteure, allié du gouvernement Monsieur Mini. Merci madame la présidente, le gouvernement tient aussi beaucoup à l'article IV qui renforce les garanties accordées aux contribuables et concourt directement à l'objectif poursuivi par le gouvernement dans le cas du projet de loi, il prévoit tout d'abord de réduire de 30 pourcent le montant du aussi de l'intérêt de retard cadre encadré Gül Ariza sont par le contribuable au cours d'un contrôle fiscal pour l'ensemble des procédures de contrôle, il vise aussi à inscrire dans la loi la procédure de rescrit fiscal en cours de contrôle et prévoit enfin que les points examinés par l'administration, lors d'un contrôle fiscal sur lesquels il a pu prendre position en toute connaissance de cause lui soit opposable, il s'agit pour nous de véritables avancées pour les contribuables, donc l'avis défavorable à cet amendement de suppression. Merci monsieur le ministre, je mets donc aux voix l'amendement 134 qui a un avis défavorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Qui quoi. Qui s'abstient l'amendement 134 ans n'est pas adopté, nous passons à l'amendement 205 présenté par le gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, je disais à l'instant, en réponse à l'amendement telle qu'il était défendu, que le gouvernement tient à l'article IV et nous tenons à ce que l'article 4 d'un article qui soit parfaitement applicable et qui permettent de mettre en place le système de la garantie fiscale dans de bonnes conditions pour que les bénéfices qui en sont attendus, soit véritablement au rendez-vous. Je disais à l'instant que cet article renforce la sécurité juridique des contribuables en rendant opposable à l'administration fiscale, les conclusions, même tacite de tout contrôle fiscal externe cette garantie ne vaut naturellement que pour des situations de faits identiques à droit constant et seulement pour des contribuables de bonne foi qui ne se sont livrés à aucune dissimulation manoeuvres odieuses cette garantie n'empêche pas l'administration, changer de position, mais du fait de la garantie, celle-ci ne vaut que pour l'avenir puisque c'est l'objet de élus il est toutefois nécessaire de clarifier le texte sur l'État reste imprécis sur le Champ sur lequel porte la garantie et cela risque par conséquent d'introduire des effets pervers, celui de pousser les vérificateurs a désinvesti des investigations toujours plus exhaustive de peur de délivrer une garantie sans avoir suffisamment approfondie, le contrôle, ce qui irait à rebours la philosophie même du texte, et celui de générer un contentieux sur l'identification des points sur lesquels porte effectivement la garantie donc pour lever toute ambiguïté sur la définition des points du contrôle pour lesquels l'administration a pris position, y compris tacitement il est proposé que le vérificateur liste les points examinés lors de ce contrôle, y compris les points les points sur lesquels l'administration a conclu qu'il ne comportait ni râleurs n'inexactitudes ni omission ni insuffisances dans le calcul des droits et taxes éligible dans la proposition rectification sur la vie d'absence de rectification pour clarifier la portée des conclusions de l'administration fiscale en cohérence l'amendement 206 du gouvernement déposé à l'article a introduit par Madame. Le rapporteur propose de modifier les articles L 49 elle 80 M de Lille, des procédures fiscales par ailleurs afin de compléter ce dispositif de sécurité juridique, il est proposé de l'appliquer également en matière de contribution indirecte et par suite de l'recodification article du Live, des procédures fiscales seul article L-80 dans le cadre d'un contrôle n'enquête en matière de contribution indirecte les points contrôlés seront mentionnés, selon le cas lors de l'information orale ou sur proposition de taxation écrite enfin cette mesure, hein, pas la même portée Sajid son examen de la situation fiscale des particuliers, les points examinés présentant souvent un caractère ponctuel, telles que la déductibilité d'une dépense d'équipement de chauffage ou les modalités d'imposition d'une prime exceptionnelle dans ces cas-là garanties prévues par cet article IV ne trouvent pas réellement à s'appliquer, alors qu'elle a en revanche tout son intérêt pour les contrôles de comptabilité des professionnels qui portent sur des points de méthode récurrents comme la durée des amortissements ou la politique des prix de transfert et c'est la raison pour laquelle le présent amendement refaire donc les juges la garantie sur les professionnels, dans le cas d'une vérification de comptable de comptabilité. En synthèse, nous apportons des précisions sur les conditions dans lesquelles la garantie est applicable pour éviter qu'il y a des imprécisions avec nos vérificateurs des vérificateurs de l'administration soit soit prise en défaut soit manque d'ambition dans la délivrance des garanties nous retirons le dispositif sur les entreprises et non pas sur les particuliers, considérant que l'intérêt réel porte sur la situation et développement des entreprises et enfin nous élargissons le dispositif au secteur des douanes, puisque actuellement le secteur des douanes et des droits indirects n'est pas inclus dans la garantie fiscale et nous proposons de l'élargir par cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre Madame Grenier avec de la commission. Merci madame la présidente serait considérés comme tacitement validé par l'administration fiscale, cela pourrait sembler la moindre des choses mais il se trouve que ce n'est pas le cas aujourd'hui, le fait qu'un vérificateur examine un point sans ne rien trouver aéro-dire ne garantit nullement d'un prochain contrôle sur les mêmes exercices aboutissent à la même conclusion la commission spéciale et très attaché à la garantie fiscale qui est sans doute la disposition la plus importante du volet fiscal de ce texte, elle est pour le coup, un véritable gage de confiance mutuelle entre l'administration et les contribuables, l'amendement du gouvernement est présenté comme un simple aménagement de la garantie fiscale les particuliers en seraient exclus, ce qui peut se comprendre, et le dispositif serait en contrepartie étendue aux contributions indirectes mais en réalité, le coeur de la mesure disparaît puisque le principe d'approbation tacite serait remplacé par un principe d'approbation expresse limité à certains des points contrôlés et à la discrétion de l'administration, la mesure serait ainsi largement vidée de sa substance par cet amendement qui supprime le principe que nous défendons, à l'issue d'un contrôle tous points examinés à condition bien sûr que ce soit en toute connaissance de cause doit être soit contestée soit validé ce que demandent les contribuables à juste titre, c'est une sortie de l'ambiguïté, donc le commentaire assez défavorable. 200 ah pardon, excusez-moi, monsieur le ministre, vous avez demandé la parole. Merci madame la présidente, madame la rapporteur ne pardonnera d'insister un peu sur les arguments du gouvernement, il ne s'agit pas pour nous de de remettre en cause le principe de la garantie fiscale juste faire en sorte qu'elle soit appliquée de la manière la plus efficace possible, vous nous rejoignez sur l'objectif de resserrer le dispositif sur les entreprises plutôt que sur les particuliers car nous avons tous conscience que c'est principalement sur les méthodes d'élaboration et les procès sur les processus récurrents que le principe même de la garantie trouve à s'appliquer, j'ai cru comprendre en tout cas pas votre film votre silence ou votre approbation tacite, pour le coup que l'élargissement aux droits indirects au secteur dédouaner quelque chose qui est aussi dans le sens recherché par la la commission spéciale de votre assemblée nous avons peut-être une divergence divergences qui est apparu et vont pardonnerai là aussi cette taquineries si j'ose dire, à l'occasion de l'adoption de l'article additionnel que vous avez proposé à la commission spéciale visant à amener le vérificateur ou les vérificateurs a dressé la ou les vérificateurs a dressé la liste des points examinés considérant par là que la liste des points examinés garantie tacite pour l'ensemble des points et en fait l'objet d'une d'une nous considérons que, en tout cas dans un 1er temps, les services de la DGSI, qui sont principalement mobilisés pour ses travaux d'inspection et de vérification devait être en capacité de lister les points qui ont fait l'objet d'une vérification en cohérence et en conformité avec les dispositions de l'amendement que vous avez proposé fait dopé par la commission spéciale mais nous considérons aussi que ce même vérificateur doit être en capacité de dire parmi les points vérifier ceux qui font l'objet de l'application de la garantie parce que ce sont ceux-ci qui ont été examinés en toute connaissance de cause et avec la garantie que le vérificateur et puis aller au bout de ses opérations de contrôle, il faut avoir en tête que dans d'autres dispositions du projet de loi que nous vous proposons et qui ont recueilli un avis favorable de la commission spéciale comme de l'Assemblée nationale, précédemment, nous envisageons de limiter la durée de contrôle que connaissent les entreprises, notamment les PME et ça ne s'appliquera par expérimentation qu'aux PME, à 9 mois sur 36, ça signifie aussi que d'une certaine manière nous avons comme objectif de réduire le temps pendant lequel ces contrôles auront lieu et que par conséquent, un certain nombre de points peuvent faire l'objet de vérifications qui, aux yeux du vérificateur ne serait pas suffisamment complète complète parfaite pour l'amener à délivrer cette garantie, et donc on a véritablement cet objectif d'efficacité effectivement passer de la garantie tacite à la garantie explicite de manière à ce que non seulement le vérificateur sont sécurisés mais aussi qu'il y ait le moins de contentieux possibles sur l'interprétation faite je suis désolé madame la prison d'avoir été un peu long mais je tenais vraiment à souligner que nous sommes attachés à ce principe de garantie, mais que la recherche d'efficacité sur ce principe de garantie, nous amène à proposer des aménagements de de l'amendement du goût Merci monsieur le ministre-ce que Madame le rapporteur Voléro prendre la parole il y a le fichier des écritures comptables dans les entreprises, donc l'administration peut prendre le fichier. écriture comptable, elle mouline en langage et elle peut sortir énormément de de points, donc je pense sincèrement qu'on peut laisser en fait, l'écriture, que nous avons de notre article ensuite. Pour effectivement le resserrer sur sur les sur les entreprises et l'élargir sur sur les contributions indirectes là à ce moment-là, vous pouvez toujours remettre dans un autre article ces ces éléments-là, mais en tout cas nous la position de la Commission, c'est toujours défavorable en fait être à votre à votre amendement bon souhaite garder l'écriture de notre article merci, cher collègue. Nous allons donc. Que passer au vote de l'amendement 205 du gouvernement qui est donc toujours un avis défavorable de la commission qui est pour.

Merci madame la présidente, le gouvernement prend acte d'une évidemment du du du vote du Sénat dans la poursuite de cette discussion sur l'article 4 et la garantie, nous avons déposé un instant et vous pardonnerez, je l'espère en tout cas cette façon peut-être un peu Cavaliere procéder à un amendement de repli, un amendement de repli qui vise dans un 1er temps et pour rejoindre un des points d'accord que nous avons à élargir le Champ de la garantie aux droits indirects et donc au secteur des douanes, de manière à ce que, au-delà de la petite divergence que nous avons, nous puissions malgré tout, à l'occasion de cette séance, faire avancer cet article sur la question des droits indirects, comme nous l'avons dit dans la défense de l'amendement 205. Merci monsieur le ministre, vous êtes en train de récupérer donc l'amendement 200, c'est ce que vient de nous faire parvenir le gouvernement, je vais demander pendant qu'on vous le distribue à Madame la rapporteure, si elle peut nous donner l'avis de la Commission sur cet amendement 216

Alors à ce moment-là, monsieur le ministre, il faut vous exprimiez parce que ça voudrait dire que l'amendement du gouvernement doit être rectifié. Monsieur miné. Merci madame la présidente, le gouvernement dépose cet amendement de repli à l'article IV car il s'agit strictement du même objet, l'article 4 défini le périmètre auxquelles s'applique la garantie fiscale et donc, par conséquent, il nous semble tout à fait logique d'ajouter la question des droits indirects dans l'article IV je ne partage pas, vous me pardonnez Madame le rapporteur, l'argument consistant à dire qu'il faudrait créer un article additionnel nous sommes sur la définition de la garantie, nous élargissons le périmètre de la garantie, conformément aux attentes, qui ont été exprimées nombreuses reprises, tant par votre commission que par un certain nombre de parlementaires à l'Assemblée et par la direction générale des douanes et les droits indirects et donc sa place logique et bien au coeur de l'article 4 qui défini le régime de garantie. Monsieur Richard a demandé la parole. et on peut pas en faire un article spécifique parce qu'il faudrait réécrire et ce qui ne serait pas préférable Monsieur le Ministre, de réserver ce là pour quelque temps, et le pouvoir, l'ajouter un peu plus tard, le temps que le service et la Commission et le temps de d'en vérifier l'impact.

La séance est reprise madame la rapporteur à vous la parole. Donc là, avec l'avis de la commission, donc nous restons sur notre position de d'être d'accord sur sur ce que voulez inscrire mais le remède dans un article additionnel. Merci madame la rapporteur monsieur le ministre. Merci madame la présidente j'entends l'argument tous quelle est la position de la Commission, mais au-delà de la conviction sur le fond que ce que nous proposons, relève véritablement Title IV et ça nous paraît devoir aller au coeur de l'article IV, il faut aussi avoir en tête une question de les justifier d'écriture législative, nous proposons un amendement. Modifié qui intervient après l'alinéa 8 de l'article IV l'alinéa 8 ayant pour objectif de modifier l'article L- 80 du code général des impôts, la proposition est la ligne à 10 qui vient juste après modifié le elle 80 B, la position que défend Madame le rapporteur consiste à introduire un article additionnel après l'article IV qui consisterait à viser une 2ème fois le elle 80 du code général des impôts, dans un article qui viendrait après l'article 4 et après que nous ayons visés au 2ème alinéa 80 et en matière, les gesticule, la logique veut et je crois que c'est reconnu et partager que les articles du code, que nous sommes amenés à modifier le soit dans l'ordre et donc dans la mesure où il s'agit d'une modification du elle nous devons introduire ces modifications par amendement avant les dispositions concernant le elle 80 B, c'est-à-dire entre l'alinéa 8 et la ligne 10 de l'article IV, c'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement sur l'article 4 à la ligne que j'ai ainsi mentionné. Donc, Monsieur le ministre madame la rapporteure, si je résume bien les choses : si vous souhaitez reprend la parole à la madame la rapporteure si la position est toujours la même : ça veut dire qu'il y a un avis défavorable de la commission. Sur l'amendement 216 heures, telles qu'il est présenté, monsieur le ministre. On veut reprendre la parole avant que je mette au revoir. Madame la rapporteur d'abord confirme sa position sert même la rapporteur : on est bien d'accord qu'un avis défavorable. Si il n'y a pas d'article additionnel. Oui, tout à fait moi je voulais juste dire du point de vue logistique qu'en matière douanière on a 3 en. Faites qui font la même chose avec les intérêts de retard donc quand vous nous dites que parce que dans l'article 4 on renvoie sur l'île des procédures douanières sincèrement on peut le faire aussi, dans un article additionnel qui vient après c'est fait dans le c'est Merci madame Bruni Monsieur le ministre. à cet endroit et c'est véritablement un principe légiste hic qui est, qui est reconnu et en terme de lisibilité de la loi et donc d'intelligibilité de la loi, y compris au regard du Conseil constitutionnel, il est extrêmement important de respecter, à notre sens, que l'Ordre des articles, nous examinons dans le code général des impôts, par ailleurs, j'appelle l'attention des uns et des autres, des sur le fait que ce que nous proposons là et après avoir pris acte de la position de la commission spéciale qui a refusé les modifications plus importantes que nous proposions de l'article IV, ce que nous proposons là va dans le sens à la fois du travail de la commission et surtout dans le sens des contribuables avec cet amendement, nous ne poursuivons Cannes, objectif : faire en sorte que la garantie fiscale qui s'applique aux impôts Directs ne soit aussi soit aussi appliquée aux impôts indirects et donc il y a une extension du Champ qui correspond parfaitement à ce que votre commission recherche et je vous invite véritablement à adopter cet amendement qui permettra aux entreprises et aux particuliers, puisque vous avez maintenu ces dispositions de bénéficier d'une garantie fiscale tant sur les impôts Directs que sur les impôts indirects, je répète, la logistique, on nous impose véritablement de maintenir à cet endroit du texte. Merci, Monsieur le Ministre, chacun a bien compris les positions, donc je vais mettre au voile amendement 200 c'est ce qui a donc un avis défavorable de la commission qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient. L'amendement n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 4 qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient, l'article 4 est adopté. Nous passons après l'article IV un amendement 28 rectifier bis. Présenté par Monsieur mouillé. Merci, présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement concerne de petites entreprises demain de moins de 21 salariés en effet en cas de procédure fiscale à la demande du comptable du Trésor, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor sous forme de cautionnement d'hypothèques de nantissement que le contribuable soit ou non en face de contentieux pour pouvoir bénéficier effectivement du sursis de paiement qui l'a demandé ces garanties sont très coûteuses pour les petites entreprises et obère leur capacité de financement cette situation conduit parfois, ça fait à choisir entre la poursuite d'un contentieux ou le développement de leur activité. Dès leur quand même que les contribuables soient de bonne foi, il est tenue de constituer des garanties lorsque celles-ci lui sont demandés de plus au terme de l'article R. 277 de duels PF et entreprises de moins de 21 salariés de bonne foi qui veut se prévaloir du sursis de paiement peut se retrouver dans une situation préjudiciable, c'est le comptable public refuse les propositions du contribuable, en effet, ce dernier se retrouvera de facto privés du droit au sursis de paiement est donc demandé et je précise bien uniquement pendant la phase de noms que de de non contentieuse une dispense totale de 10, constitution de garantie en cas de sursis de paiement. Merci, cher collègue, avis de la commission Madame Bruni-. Merci, même la présidente. Pour la Commission, c'est une demande de retrait, alors on est bien conscient que constituer des garanties, ça peut être difficile voire très difficile pour un redevable qui sollicite un sursis tellement ceci dit supprimer cette obligation ferait courir un risque trop important au Trésor public, bien sûr, mais surtout à l'entreprise elle-même si la réclamation venait à être rejeté, au final, cette disposition risquerait d'aboutir à une hausse des défaillances d'entreprises plutôt que l'inverse alors je rappelle toutefois que les garanties ne sont pas nécessairement constitué en espèces peut s'agir de marchandises de titres ou encore d'une caution bancaire, c'est peut-être d'ailleurs là que se trouve la solution au problème posé par votre amendement l'accès des TPE et PME auprès et caution bancaire et là je j'ai une question pour monsieur le ministre est-ce que le gouvernement a l'intention de traiter ce problème dans le cas de la loi pacte annoncé pour cette année. Merci madame la rapporteur, Monsieur le Ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présidente sur sur l'amendement qui vient d'être présenté là l'avis du gouvernement est le même que l'avis de la commission, ce qui me demande de retrait pour les mêmes arguments et à défaut, un avis défavorable, pour ce qui concerne la question des des cautions, vous avez évoqué, vous savez que la phase la loi pacte est encore dans une phase de consultation de concertation, le texte n'a pas encore été transmis au Conseil d'État n'a pas encore été examiné par le Conseil des ministres, donc il encore dans l'élaboration et la proposition vous faites sera évidemment transmise à nos collègues du ministère de l'Économie, des Finances, quelles mesures il pourrait intégrer ou pas, ces dispositions dans le texte prépare. Si Monsieur Bouillet. je vais retirer l'amendement, puisque non pas : nous avons une garantie de la part du ministre, en tous les cas une garantie de transfert ou de en tout cas de discuter de ce sujet le cas contraire je sera représentés dans ce texte-là, mais il n'empêche que, au regard de l'argumentaire comme je ai bien précisé que cet amendement porte principalement lorsqu'on n'est pas en face de contentieux je comprends tout l'argumentaire lorsque le ensuite enclenché la nécessité de pour l'entreprise et pour les années public de faire ses ses provisions, mais lorsque le contentieux n'est pas engagé, on ne sait même pas ce que volet et donc je pense que cette nuance pouvait justifier un avis favorable de la commission, j'entends ces éléments mais il n'empêche que nous serons extrêmement vigilants lors des prochains débats dans les semaines qui viennent, donc je retire l'amendement. Merci, cher collègue, l'amant ment 28 rectifier bis s'est retiré.

oui. Le président peut nous administre alors le présent amendement vise à appliquer le principe du droit à l'erreur, promu, notamment en matière fiscale par le projet de loi à la mise en 9 du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, l'amendement propose qu'à compter de 2019, et pour les 2 premières années suivant celle de l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et les personnes physiques, en charge du traitement ne soit pas redevables en cas d'erreur à l'obligation d'effectuer la retenue à la source des pénalités prévues à l'article 1759 0 A du code général des impôts, si leur bonne foi et reconnu. à ce jour d'ailleurs, notons que à ça tombe d'entreprises n'ont pas répondu l'obligation concernant les déclaration sociale nominative qui est assigné et donc un risque de difficultés à venir, le rapport de l'IGF d'ailleurs pointe ces mêmes difficultés et avait aussi proposé l'instauration d'un si le droit à l'erreur, voilà donc le jet de cette amendement. Si Monsieur mouillé, l'amendement 186 rectifier lycées présentée par Madame Nathalie Delattre. Oui, madame la présidente, je pourrais dire qu'il est défendu mais je rajouterai effectivement que ce prélèvement à la source, sans impose aux entreprises, c'est vrai que c'est un moment très anxiogène, puisqu'elles ont énormément de de questions, elles seront aussi questionné par les salariés qui auront beaucoup de de problématiques et de questionnement, ils auront d'ailleurs des réticences, a appelé l'administration parce que ce sera en appel le j'en parlerai puisque j'ai eu un amendement il recevable sur l'article 15 mais effectivement, ce n'est pas de nature à rassurer et si le gouvernement pouvait accepter cet amendement qui permettrait aux entreprises de pouvoir de moins de 150 salariés de pouvoir aborder ce grand saut dans l'inconnu, serait effectivement une preuve de confiance. Collègues nous passerons à la présentation par monsieur toujours de l'amendement 30 rectifier bis. Oui, mais le président, Monsieur le Ministre, alors cet amendement est plutôt un amendement de repli qui diminue donc le le la, la, la base à moins de 21 salariés

sur sur le de 33, ce sera une demande de retour. Et sur le 186 également et le 30, un avis favorable alors qu'on sait très bien que de nombreuses PME rencontre des difficultés dans la préparation du prêt prélèvement à la source et en amont de la déclaration sociale nominative d'ailleurs Monsieur le ministre, à priori, il reste encore 30000 petites entreprises qui n'ont pas encore intégré la déclaration sociale nominative dite DSN que ce soit pour la DSN pour ces petites entreprises ou pour le prélèvement à la source, j'espère que l'État sera bienveillant parce que l'État nous a quand même demandé de repousser, c'est justement sur l'application de la DSN pour son administration, donc ça on vous demande vraiment un un engagement à ce sujet, voilà, alors il n'est cependant pas raisonnable de supprimer purement et simplement les pénalités applicables pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés ne s'agit pas uniquement de PME et pour les plus grandes, la mise en oeuvre du prélèvement à la source devrait soulever moins de difficultés, et si cette amendement était adopté alors les entreprises qui n'encourt plus aucune sanction attendraient le dernier moment et demanderaient un délai supplémentaire, comme le fait l'état, d'ailleurs, nous nous retrouverions avec le même problème, 2 ans plus tard, des scènes d'ailleurs a eu plusieurs fois des délais supplémentaires, donc nous acceptons bien entendu le le seuil de 21 salariés parce qu'effectivement, les très petites entreprises, ils ont beaucoup de mal à appliquer ces nouvelles dispositions ensuite pour répondre à Madame Delacroix qui s'inquiète effectivement des questions des des salariés, hé bien moi je pense que les salariés, il faudra les envoyer vers l'administration parce que, effectivement, effectivement, dans les entreprises, ça va poser un problème et pas seulement sur des questions mais aussi sur cette agression sur leur bulletin de paye parce que, comme pour beaucoup de salariés regarde surtout le bas du bulletin, ils vont se sentir agressés dès le bulletin de paie du mois de janvier, en pensant que leur entreprise à diminuer leur salaire d'certainement une ambiance aussi dans les entreprises qui sera beaucoup plus difficile, voilà donc demande de retrait, donc sur les 2 premiers amendements et sur le tremplin, un avis favorable, madame la présidente. Merci madame la rapporteur, Monsieur le Ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présence d'un débat que nous avons eu en commission, y compris, et lors de l'examen des articles et en fait l'objet d'une approbation d'une adoption pardon par la la nouvelle procédure législative et qui avait aussi été menée dans le cas des débats à l'Assemblée nationale, un justement de d'amélioration du dispositif ont été adoptés, le gouvernement avait reporté d'un an la mise en eau du prélèvement à la source justement pour garantir les meilleures conditions techniques d'efficacité, de mise en place du dispositif et il faut rappeler que pour répondre aux craintes exprimées par les collecteurs et tenir compte des recommandations formulées par la mission d'audit de l'IGF, l'article 11 de la 2ème loi de finances rectificative pour 2017 a déjà réduit de moitié en passant de 500 à 250 euros le montant minimal de l'amende applicable en cas de défaillance déclarative du collecteur en août, le gouvernement a accepté lors de la dernière loi de finances rectificative pour 2017 n'a proposition d'alléger les sanctions pénales auxquelles rétention de la retenue à la source, s'inspirant notamment des dispositions qui existent en matière sociale par rapport au dispositif initial, c'est déjà un ajustement important par ailleurs pour répondre à Madame la rapporteure, la ligne de conduite de l'administration fiscale sur celle qu'elle suit chaque fois que sont mis en grève, de nouvelles réformes d'envergure comme l'introduction des déclarations préremplies : lancement de la télédéclaration la généralisation des télé-procédure aux petites entreprises, à savoir un simple rappel des obligations applicables sans appliquer de sanctions pour les premiers mois de manière à ce que la pédagogie puisse être faite avant qu'il y a sanction enfin dans le cas de la mise en oeuvre, pour la première fois d'une réforme d'ampleur comme celle du prélèvement à la source, qui implique une bonne mobilisation particulière des collecteurs, au risque de menacer la collecte d'impôts, il faut aussi préserver le cadre dans lequel les choses sont effectués et le maintien d'un régime de sanctions même allégé même aménagé, même avec une disposition transitoire est utile à l'efficacité et à la réalité de la mise en oeuvre, j'ajoute un mot si vous le permettez, parce que nous avons d'échange en commission spéciale pour dire que le gouvernement travaille avec la société des éditeurs, des bulletins de paie et que nous avons eu l'occasion de rencontrer, j'ai participé à leurs travaux d'assemblées générales en début d'année, une charte a été signée tout récemment entre l'Inde et j'ai Philippe et la société des éditeurs pour permettre une diffusion et une généralisation de systèmes d'édition de pays qui intègre les modalités nécessaires au prélèvement à la source, et nous avons par ailleurs travailler avec cette société des éditeurs pour faire en sorte que pour celles et ceux des entreprises, des chefs d'entreprise, pardon, et donc des pour celle des entreprises qui sont équipés de logiciels relativement récent, et notamment ceux qui sont équipés en déclarations sociales nominal nominative Lise l'introduction des éléments nécessaires au prélèvement à la source soient imputés sur les charges de maintenance et non pas considéré comme un investissement nouveau de manière à ne pas amener ces entreprises à payer 2 fois, des investissements en matière d'édition ne paye une fois il y a quelques mois pour la décennie et qu'il sera amené à renouveler pour le passe, donc nous travaillons avec associe des éditeurs pour aller dans le sens que vous appelez de vous.

Juste par rapport à ce que vous venez dire Monsieur le le ministre concernant effectivement cette négociation avec les les éditeurs pour que le prélèvement à la source soit imputée sur la maintenance informatique, donc bien entendu, je vous remercie de l'avoir rappelé, j'allais vous le demander, en revanche, ce qu'il faudra essayer essayer de faire, c'est d'en faire la publicité auprès des entreprises, parce que les éditeurs, on peut leur faire peut-être confiance puisque nous sommes ici dans un climat de confiance, mais elle est toute relative, voilà merci beaucoup.

Oui pour dire d'abord à la présidente que je crains que les salariés des réticences, le administration parce que comme je vous le disais, ce sera un appel surtaxé donc les chefs d'entreprise auront malheureusement devoir répondre à des questions qui ne concernent pas vous dire que nous retirons au jour retire le 186 rectifier pour voter la demande non présenté par Monsieur. Merci, cher collègue, le 186 rectifier Bissey retiré et nous allons mettre on voit l'amendement 30 rectifier bis qui a été présenté par Monsieur mouillé qui est pour. Qui est commun. Qui s'abstient l'amendement 30 rectifier bis est adopté article 4 bis à nous avons un amendement 135 qui est présenté par Monsieur Oui merci ne la présidente un article ajouté en commission qui n'apporte pas, selon nous, de de réelle plus-Value, le texte de l'article L-49, issu de la loi de finances rectificative pour 2016 promulguée il y a moins d'un an et demi était selon nous suffisamment explicite quelle effectivement la plus-Value cet article du point de vue du contribuable pourquoi alourdir le texte de l'article 49 du livre des procédures fiscales en lui ajoutant les références d'autres articles dont le contenu est moins générique et plus concret, ayant par conséquent le défaut récurrent d'une excessive précisions à l'article 49 est simple, il traduit la volonté du législateur d'indiquer dans la relation entre l'administration fiscale et le contribuable. Que celui-ci est en droit de recevoir un document établissant les résultats des contrôles effectués merci. Si madame la présidente, cette disposition est de nature à créer un un climat de confiance entre les entreprises et l'administration et n'est pas redondant par rapport au droit existant en effet les prises de position formelle de l'administration lors d'un contrôle fiscal sont des facto limitée au point faisant l'objet de réhaussement et qui figure sur la proposition de rectification, le fait que le vérificateur ne propose pas de rectification sur les autres points examinés ne signifie nullement qu'il considère ceci comme conforme à la loi fiscale dès lors ces points sont susceptibles d'être remis en cause en cas de contrôle fiscal ultérieures et portant sur les mêmes exercices ce qui est source d'insécurité juridique pour les entreprises, avec cet amendement, le contribuable serait expressément informé des points que l'administration considère comme conforme à la loi fiscale et il nous semble, c'est la moindre des choses, alors que le gouvernement appelle à davantage de confiance et de transparence. Donc défavorable. Merci madame la rapporteur, Monsieur le Ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présidente, j'ai eu l'occasion de dire précédemment que cet article 4 bis qui est né d'un article additionnel adopté par la commission à l'initiative de Madame rapporteur était un article que j'ai recueilli la sonde seulement du gouvernement, que nous aurions préféré que le la liste des points faisant l'objet d'une garantie soit une liste explicite pour ne pas refaire le débat que nous avons, il y a un instant, mais il n'empêche qu'en l'état et à ce stade des discussions, le gouvernement a toujours favorablement de son âge relocation proposés dans un instant des amendements de coordination à cet article donc par conséquent nous sommes défavorables, sa suppression. Merci, Monsieur le Ministre, donc nous allons mettre aux voix l'amendement 135 avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté, amendement 206 présenté par le gouvernement Monsieur mini. Merci madame la présidente, d'espèces, je ne désespère jamais de convaincre, d'élargir le Champ de la garantie aux droits indirects et la direction générale des douanes l'amendement 205 ils ont été rejetés, ainsi que l'amendement 216 la maman de sens 206 n'a plus de sens, il est retiré. Merci monsieur le ministre, l'amendement 206 s'est retiré, je vais mettre aux voix l'article 4 bis à qui est pour. Qui quand même. Qui s'abstient, l'article 4 bis est adoptée après l'article 4 bis à un amendement 212 présentée par Madame Bruni au nom de la commission spéciale. Merci madame la présidente, alors qu'elle était courantes avant la mise en place du bulletin officiel des finances publiques, le beau philippin 2012, la publication des rescrit est aujourd'hui très occasionnel, alors qu'elle contribue à la sécurité juridique des contribuables et qu'elle réduit le risque de contentieux lors de son audition par la commission spéciale, le directeur général des finances publiques a reconnu qu'un effort en la matière était nécessaire, toutefois, la décision de publier les rescrit demeure aujourd'hui entièrement discrétionnaire et seule une part très réduite 18000 rescrit traitées chaque année et rendue publique, les prises de position formelle, sa situation spécifique d'un contribuable ne sont pas concernés par l'amendement et ne seront donc pas publié. Merci madame la rapporteure, monsieur le ministre, Merci madame la présidente, le gouvernement partage la la volonté de la rapporteure de voir publier les rescrit qui ont une portée générale, si j'ai l'occasion de le dire devant votre commission, comme d'ailleurs publiquement à l'occasion de déclarations dans la presse, la direction de la législation fiscale et le service juridique de la DG Philippe ont pour pratique de publier les clarifications utiles à la bonne compréhension des règles en vigueur nous considérons qu'il faut aller au-delà, en relançant la publication des rescrit sous forme anonymiser, bien entendu, de manière à donner rose entreprises aux particuliers, des exemples concrets illustrant l'application de la règle fiscale pour autant, il n'apparaît pas utile au gouvernement de légiférer pour atteinte cet objectif je prends à nouveau l'engagement devant vous au nom du gouvernement de développer la publication des rescrit généraux cette publication fait partie des consignes données la déjà Philippe pour améliorer l'information des contribuables sur les récuse qu'elle s'applique à leur situation et je peux vous annoncer madame la rapporteure la création dans les prochaines semaines d'une base des rescrit justement pour généraliser généralisée et amener nos services publié plus fréquemment plus régulièrement les réinscrit à caractère général que vous le demandez par cet amendement considérant véritablement que légiférer nous paraît excessif, qu'il faut qu'il y a aussi une possibilité d'appréciation par contre la généralisation de la procédure et la création de la base de nous permettent d'être beaucoup plus efficace en la matière et je le répète, un engagement pris devant vous.

rêve bien madame la rapporte. Auteur, donc je vais mettre aux voix l'amendement 212 de la commission spéciale qui est pour.

Merci madame la présidente, monsieur le ministre, cet cet amendement de notre groupe participent quelque peu des mêmes par l'ONU, les mêmes observations que celle que vous avez pu produire sur l'article précédent et l'amendement 135. et elle 13 j'ai du Live, des procédures fiscales portent d'une part sur les procédures de vérification générale de compèt de comptabilité dans le cas d'un contrôle sur place, d'autre part sur les procédures d'examen de la situation fiscale personnelle et enfin les procédures de contrôle de compèt de comptabilité informatisée par voie télématique, ce qui signifie que l'ancienne, l'essentiel des procédures de contrôle fiscal externes qui sont en quelque sorte le dur du travail de contrôle fiscal sont placés hors Champ d'application du présent article il sait gérer, donc de donner une qualité nouvelle recours expédiés à l'endroit d'un supérieur hiérarchique immédiat ou non d'un vérificateur, mais le tout dans le cas d'une procédure qui n'est pas la plus traumatisante en oubliant pas que l'article 54 B. du Live, des procédures fiscales, indique pour sa part, je cite la notification d'une proposition de rectification doit mentionner sous peine de nullité que le contribuable à la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre, nous avons donc avec cet article, rien d'autre qu'un encouragement à la mise en oeuvre d'une manoeuvre d'attente dont les conséquences pourraient d'ailleurs s'avérer contre-productive, et dont l'un des effets pourraient être d'inciter l'administration à réaliser un examen de contrôle plus approfondi que celui découlant d'un simple contrôle sur pièces, une telle démarche en durcissant inutilement des procédures contentieuses limité, va sans doute à l'compte de l'instauration d'une relation de confiance entre l'administration et usagers, nous ne pouvons donc vous inviter à adopter la suppression de cet article, merci. Merci monsieur Gontard Madame Bruni, avis de la commission. Merci madame la présidente, ce sera un avis défavorable, c'est exactement ce qui existe actuellement en matière de contrôle sur place, donc c'est une garantie supplémentaire qui offerte aux contribuables qui devrait contribuer à améliorer le dialogue avec l'administration dans la phase pré-contentieuse et à réduire ainsi le nombre de contentieux je précise enfin que cette voie de recours serait exclue pour les procédures de taxation d'office réservée à des contribuables qui ne s'acquittent pas de leurs obligations défauts déclaration l'absence de réponse à une demande de l'administration et l'opposition a contrôle fiscal, donc c'est vraiment d'adapter les mêmes mesures, les mêmes possibilités que ce soit un contrôle sur place pour un contrôle sur pièces, donc un avis défavorable pour cet amendement. Merci madame la rapporteur, Monsieur le Ministre à vie du gouvernement.

Qui s'abstient l'amendement 136 n'est pas adopté, je mais au voile article 4 bis qui est pour. qui est pour. Qui. Qui s'abstient, l'article 4 bis est adoptée article 4 terre amendement 176 rectifié présenté par Madame de la. Oui merci madame la présidente, cet article, introduit à l'Assemblée Nationale prévoit l'accès au public des informations détenues par l'administration fiscale relative aux valeurs foncières à l'occasion de mutations intervenues au cours des 5 dernières années, je souhaitais simplement signaler que depuis la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique cet accès a été largement partagé notamment par des personnes publiques ou privées, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences ou de leur activité, tels que des chercheurs, des activités de services contribuant à l'information des vendeurs et des acquéreurs des établissements publics des agences d'urbanisme sérénades SFR des professionnels et beaucoup d'autres et des particuliers ayant un intérêt à consulter ses données, je trouve que il n'a pas été suffisamment motivé l'intérêt de rendre une totale prend transparence à l'ensemble effectivement qui ne sont pas forcément demandeurs de cette mesure et on sait que ce sont des risques de de confidentialité qui peuvent être porteurs de problématiques, donc voilà, nous proposons de supprimer cet article.

parce que faut-il vraiment rendre accessible à tous sur internet des données telles que l'adresse, la surface et le prix de vente des biens immobiliers, alors en vérité, c'est effectivement ce service existe déjà : il s'agit, il s'appelle Patrimoine il est disponible sur impôts Point la différence c'est qu'il faut aujourd'hui s'identifier et justifier d'une raison valable pour consulter ces informations notamment en vue d'une vente ou d'une acquisition, par exemple, la commission a adopté plusieurs amendements pour encadrer strictement le nouveau dispositif et garantir la protection de la vie privée en excluant toute identification nominative des propriétaires des biens et en prévoyant un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ni claques ni alors il me semble que cette approche est préférable à une suppression pure et simple de l'article qui risqueraient sinon d'être rétabli dans sa version initiale, par l'Assemblée nationale pour information cet article avait déjà eu. Adopté dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2017, mais elle avait été censurés comme cavaliers législatifs, par le Conseil constitutionnel, donc c'est plutôt une demande de retrait sinon un avis défavorable. Si Madame la rapporteure avis du gouvernement Monsieur Mini-. Merci madame la présidente, madame Delattre a rappelé que depuis la promulgation de la loi pour une République numérique, il y avait déjà une seconde d'obligation à l'Assemblée nationale a voulu justement répondre. Et une difficulté d'accès aux données prévue par la loi pour une République numérique, accès pour les uns et les autres, vous avez d'excès pour tout ça que c'est aussi d'ailleurs pour les collectivités ou les aménageurs qui ont besoin des informations pour mener à bien leur projet et par l'ARC, la banque adopté par l'Assemblée, ces difficultés était levé, la commission spéciale du Sénat a souhaité renforcer les obligations d'anonymisation des données qui sont fournis, au-delà du seul nom des propriétaires tels que c'était prévu des dispositions adoptées à l'Assemblée nationale l'article telle qu'il est sorti de la commission spéciale convient parfaitement au gouvernement et donc nous souhaitons le maintien, c'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à sa suppression et que nous vous demandons le retrait de cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre, que fait Madame de la. Oui au retrait confirmé. Alors l'amendement 176 et rectifier et retiré je mets donc on voit l'article 4 qui est pour.

merci de la présidente celui chers collègues notre amendement relatif au droit à l'erreur en matière douanière droit qui est d'ailleurs déjà existants, reprend pour une part essentielle des termes prévus par le texte du projet de loi lui-même, s'agissant du droit à l'erreur, de manière générale, il s'agit donc de faire en sorte que les critères d'atteintes à l'environnement à la sécurité, à la santé publique, ainsi que les infractions touchant de dispositions fondamentales et d'ordre public, du droit du travail soit retenu pour exemple l'application du droit à l'erreur, guillemets, notre souci est donc un souci de logique et de cohérence du texte, s'agissant du droit à l'erreur en matière douanière de la faculté de transiger, l'article 350 du code des douanes fixe clairement les règles de ces transactions, il existe donc d'ores et déjà une grâce une graduation clair de l'action publique et de la faculté de transiger dans le domaine douanier. Merci madame la présidente, ce sera un avis défavorable, l'article 4 quater permet de réduire l'intérêt de retard de 50 pourcent en cas de régularisation spontanées de 30 pourcent cadre aiguë arrestation au cours de contrôle pour les droits et taxes recouvrer sur le fondement du code des douanes, en excluant les régularisations portant sur des produits liés à la santé, à la sécurité à l'environnement en droit du travail aux normes internationales votre amendement viderait largement de son sens le dispositif, alors ce n'est pas justifiée, on peut commettre une erreur de bonne foi, quel que soit le type de produits concernés puisque c'est une erreur et la réduction des intérêts Dreux retard ne s'applique qu'à condition que le contribuable bien sûr soit de bonne foi et qu'il régularise son erreur, donc pour les déclarations volontairement et la réduction des intérêts de retard n'est de toute façon pas possible et les sanctions sont pleinement applicables. Et merci, merci, madame la rapporteur, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, l'avis est défavorable pour pour les mêmes raisons, j'ajoute que, en la matière, les régularisations concernés portent sur la fiscalité énergétique ou environnemental sur la taxe à l'essieu et dès lors, les conditions supplémentaires, vous proposez concernant des produits portant atteinte prévu ça sur la santé publique, la sécurité des personnes et des biens, ou encore la protection d'environnement, le respect des normes internationales ne nous paraissait pas pertinent tué gare régularisation visés par l'article, donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci, je mets donc aux voix l'amendement 137 qui a un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. qui est pour. Quand. Qui s'abstient l'amendement 137 n'est pas adopté, nous passons à l'amendement 40 présenté par le gouvernement Monsieur le ministre. Amendements rédactionnels avis de la commission. Asie favorable : avis favorable de la commission sur l'amendement 40, je le mets au voix qui est pour.

qui est pour. C'est quoi. S'abstient, l'article 4 quater est adopté article 4 Khimki s'2 amendements identiques de suppression faisant l'objet d'une discussion commune. Tout d'abord relais amendement 41 qui est présenté par le gouvernement Monsieur mini. Merci madame la présidente, l'article IV qui inquiète du présent projet de loi prévoit pour l'application de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, dite du travail d'une d'une part que le contribuable ne soit tenu d'envoyer à admis à l'administration de la déclaration annuelle de suivi de son engagement de conservation des titres question mise en demeure de l'administration et, d'autre part c'est exonération partielle ne soit pas remise en cause parce que les pièces justificatives exigées y compris autre que cette déclaration annuelle sont produits dans un délai d'un mois sur une mise en demeure par l'administration, nous considérons que cette disposition n'a pas sa place dans le projet de loi, il en est, il a en effet annoncé, le gouvernement a en effet annoncé, pardon, dans le cas du plan d'action pour la croissance et transformation des entreprise son intention de proposer, dans la perspective du projet de loi finance pour 2009 2019, des mesures fiscales qui tend. Qui tendent à favoriser davantage la transmission d'entreprise, dans ce cas, ne pourront être amenés à proposer au Parlement un assouplissement des obligations déclaratives associée au dispositif, et nous sommes préférable d'envisager globalement l'ensemble des mesures touchant dispositif du travail lors de l'examen parlementaire en loi de finances et ses propositions, c'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de l'article IV qui inquiète.

Merci madame la présidente, monsieur Ministre, mes chers collègues, hé bien oui, nous voici en présence d'un amendement déposé par notre groupe qui était identique à celui proposé par le gouvernement, j'avoue que c'est un plaisir mais une fois n'est n'est pas coutume c'est vrai que il s'agit, il faut le souligner d'un article du Code général des impôts, le 787 B relatifs au traitement fiscal des engagement collectif de conservation profondément modifié par la loi de finances pour 2018 et objet d'une nouvelle réécriture la semaine dernière dans le cadre de l'examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit des sociétés, si le gouvernement est cohérent avec la position exprimée par le présent débat il importerait qu'il procède à la suppression de l'article de cette proposition de loi, si elle vient en seconde lecture à l'Assemblée avant la fin du parcours législatif du présent texte dont nous n'allons pas faire de longs discours, mais simplement relevé le 787 a a beaucoup perdu de sa raison d'être, avec la disparition de l'impôt de solidarité sur la fortune dont il a pu constituer l'un des correctifs, alors il est temps de supprimer cet article 4 qu'inquiet, c'est de rendre ce projet de loi un peu plus intelligible car on peut tout de même se demander en quoi l'administration accompagne quant à l'adresse des mises en demeure à l'endroit des administrés, je vous remercie. Si Madame avis de la Commission sur ces 2 amendements. ce sera un avis défavorable, alors pour bénéficier du dispositif du travail sur la transmission d'entreprise familiale, les repreneurs doivent transmettre chaque année une attestation qui certifie qu'il conserve toujours les parts de l'entreprise, le simple défaut de transmission de cette attestation suffit à faire perdre le bénéfice du pacte Dutreil ce qui apparaît complètement disproportionnée au regard du manquement l'article 4 qui a une pièce adopté par la commission spéciale permet de conserver le bénéfice du pacte Dutreil si l'attestation fournit dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'administration, c'est une mesure pour nous de bon sens à équilibré et surtout cohérentes avec l'esprit du projet de loi parce que le là on est vraiment dans un cas de droit à l'erreur, alors, d'après le gouvernement, effectivement elles existe en pratique une tolérance en cas de retard mais il semble que celle-ci ne soient pas uniformément appliquée appliquée sur le territoire français, alors l'inscription dans la loi permettra de régler ce problème, il s'agit vraiment d'une simple mesure de procédure qui n'est pas du tout lié à la réforme de fond du dispositif qui effectivement promise par le gouvernement dans le cas de la loi pacte, c'est vraiment le cas du droit à l'erreur de Lublin, envoi d'une attestation donc défavorable. Merci madame la rapporteur monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci madame la présidente, pour préciser que le gouvernement maintient l'amendement de bord parce que, comme le rapporte rappeler Madame la sénatrice, la chose n'est pas forcément commune mais depuis le début de cette séance, nous citons en permanence une citation célèbre Reims, rappelons que la confiance n'exclut pas le contrôle, donc, à force de la cité, ce type d'alliance devait aussi maître dans l'hémicycle par ailleurs et pour revenir au fond, je répète à l'attention de Madame le rapporteur, que nous préférons nous préférions largement pouvoir examiner l'intégralité des dispositions relatives au dispositif Dutreil à l'occasion de la loi Paris et la votre finance qui suivra, plutôt que de prendre le risque d'insérer des dispositions dans ce texte, avec un problème aussi de lisibilité sur les dispositions qui seront progressivement prise dans cette année. Si Monsieur le ministre, je mais maintenant on voit les 2 amendements identiques de suppression. Qui ont reçu un avis défavorable de la commission qui est pour.

merci la la présidente ce mini-chers collègues ainsi que de l'avons avons eu l'occasion de le dire lors de la discussion de l'autre amendement 137 le droit à l'erreur existe de longue date, autant en matière fiscale ou il procède quasiment de l'activité quotidienne et services qu'en matière douanière, il est même codifié dans le cas de l'article 350 du code des douanes, je n'ai pas cité ici parce qu'il serait un peu long, chacun l'a bien sûr en tête, on pourrait d'ailleurs estimé que le code des douanes propos ce que pourrait être une préfiguration de l'importance donnée au droit à l'erreur et à la bonne foi des contribuables mais on aura noté que l'article 350 laisse effectivement dans certaines limites toute latitude aux services déconcentrés pour appliquer la loi avec mesure et que les recours hiérarchique découle naturellement de l'importance de la fraction à telle à telle point qu'un document syndical dont nous avons eu communication, dans le cadre de la préparation de l'examen de ce texte, nous indique, je cite en matière douanière, l'article 350 du code des douanes prévoit la possibilité pour l'administration des douanes de transiger, cette transaction a pour effet d'éteindre l'action pour l'application des sanctions fiscales, douanières, ainsi que l'application des peines d'emprisonnement prévues par le code des douanes, il convient ici de rappeler que les infractions font l'objet d'une transaction dans 99 pourcent des cas qu'elle aboutisse dans 20 pourcent à la suppression totale des de citation nous sommes donc avec cet article 600 présence concrète dans la valeur ajoutée ne mérite même pas d'être prises en compte, nous ne pouvons donc confirmer que nous ne voterons pas. Merci, Monsieur Bocquet. Nous passons à la présentation par le gouvernement de l'amendement 43. Merci madame la présidente, simplement pour rappeler que le droit à l'erreur, permet de ne pas appliquer les sanctions prévues par le code des douanes lorsque le redevable de bonne foi, rectifie de manière spontanée avant l'expiration du délai relatif au droit de reprise de 3 ans de l'administration, une déclaration qu'il à souscrites ou alors qu'un contrôle de l'administration des douanes est en cours, les les n'inexactitudes l'omission d'insuffisance a été commise, pour la première fois au cours du délai de prescription de la poursuite de l'infraction, pour ce qui concerne cette infraction commise de bonne foi, le délai de prescription et conformément à l'article 351 du code des douanes de 3 ans dans la main, dans la mesure où l'article 6 prévoyait un délai de 6 ans, les précisions combien de remplacer une décision par 3 ans de manière être en conformité avec le délai de prescription. Si Monsieur le Ministre, avis de la commission. Madame Bonino. Oui, madame la présidente, c'est un avis favorable. Favorable de la commission Genèse voilà Mandement 43, qui est pour.

Merci madame la présidente, réduit la définition du détournement de destination privilégiée la combinaison, constate la constatation d'un usage du produit que celui que vous droit à une fiscalité privilégiée et à l'absence de justification de cet usage aujourd'hui ces conditions ne sont pas cumulative et permet de prendre en compte des situations où un usage non conforme à celui qui voulait droit une fiscalité avantageuse, a pu être constaté et celle où, après que le produit qui a bénéficié d'une fiscalité avantageuse, a été consommé les services prouve qu'aucun des justificatifs, témoignant d'un usage ouvrant droit à une fiscalité avantageuse n'existent en réalité les gens les enjeux fiscaux recouverts par ces régimes sont importants puisqu'il s'agit d'une dépense fiscale de 5 9 milliards d'euros justifier suivi de ces derniers jusqu'à leur utilisation finale ouvrant droit au taux réduit ce suivi d'ailleurs similaire à celui qui s'applique à d'autres régimes d'exonération de TCP, les distributeurs doivent effectuer le suivi des produits que leur livraison utilisateur l'utilisateur doit quant à lui s'identifier auprès de son distributeur et justifier la destination des produits auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, l'utilisateur est responsable de tout usage différent de celui prévu par régime privilégié dans le cas du Caire, il acheter ces produits, la répartition des responsabilités entre distributeurs et utilisateurs est ainsi cohérente et indispensable pour assurer une traçabilité jusqu'à l'utilisation, et donc pour toutes ces raisons, demandons le rétablissement de l'article 265 B du code des douanes. Merci monsieur le ministre madame la rapporteure. aujourd'hui les distributeurs de carburant sous condition d'emploi gazole non routier agricole et fioul domestique peuvent faire l'objet d'un redressement fiscal s'ils ne sont pas en mesure de présenter le justificatif de destination des produits vendus et cela même si aucun détournement n'est avéré, ou même s'ils ne sont ni complice ni informé du détournement en supprimant l'article 6 bis adopté par la commission spéciale, nous reviendrions donc à une situation où les sanctions peuvent être disproportionnée par rapport au manquement, alors même que les distributeurs sont de bonne foi, je suis donc défavorable à l'amendement du gouvernement, ceci dit, les distributeurs sont tout de même responsable du suivi des produits jusqu'à leur destination et il n'est pas anormal de leur demander bien entendu un justificatif mais plutôt que de supprimer plus purement et simplement cet article Monsieur Münich, faudrait peut-être travailler à une solution intermédiaire, alors peut-être pour après, pour la Commission mixte par exemple sous la forme d'une amende forfaitaire en cas de non-présentation du justificatif, ce qui permettrait de maintenir quand même des sommes qui pourraient être acceptables en cas de manquement de de l'entreprise, mais pour le moment nous sommes défavorables à la suppression de cet article. Merci madame la rapporteure, je vais donc mettre aux voix l'amendement 44 avec un avis défavorable de la commission qui est pour.

madame la présidente, monsieur le ministre, nous proposons la suppression de cet article d'habilitation pour plus plusieurs raisons au-delà de position d'opposition de principe à l'application de l'article 38 utiliser plus de 500 fois durant le quinquennat précédent et déjà invoqué à 40 reprises depuis le début du quinquennat actuel singulièrement parce que le sujet est d'importance et qu'il ne saurait être limité à un dialogue entre le gouvernement et les milieux de l'entreprise, il s'il s'agit de la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux autant dire toutes les entreprises et de les mettre en situation de bénéficier d'une forme d'extension du rescrit fiscal questions déjà traitées ces dernières années pour rappel, quelques points, le délai d'habilitation ouvert et de 9 mois, ce qui, pour peu que l'on veuille ordonnances concernées nous amène, au-delà du 31 décembre 2018, de fait, alors que la procédure fiscale est un pur objet de discussion d'une loi de finance ou d'une loi de finances rectificative nous allons placer les des entreprises en attente d'application d'un cas d'législatif qui pourrait être défini tranquillement par la discussion budgétaire s'il s'agit par ailleurs de fixer des principes d'interventions des services déconcentrés et des directions spécialisées d'administration fiscale, soulignant que les faits sont déjà établis et que les plus grandes entreprises constitue déjà la clientèle privilégiée de la Direction des grandes entreprises, les PME et TPE constituant les sujets d'intervention des services territoriaux le partage existe déjà et n'est d'ailleurs pas sans poser de problème puisque la qualité du contrôle fiscal, par exemple, dépend beaucoup de l'efficacité et du travail du réseau de finances publiques à la base, n'oublions pas pour prendre un exemple en matière de fiscalité personnelle que l'affaire Cahuzac fut d'abord le résultat du travail d'un inspecteur des impôts, travailleur dans le centre des impôts de Villeneuve-sur-Lot, le gouvernement aurait mieux fait de proposer un texte de réécriture partielle du code général des impôts, plutôt qu'à Martigues d'habitation qui va priver le Parlement d'un débat pourtant utile, merci. Merci madame la présidente, ce sera un avis défavorable à la relation de confiance qui consiste à accompagner les entreprises en amont de leurs obligations déclaratives, c'est-à-dire dans une démarche de validation a a priori plutôt que de contrôle a posteriori est un élément important du projet de loi auquel la Commission spéciale est attaché, en l'espèce l'habilitation apparaît nécessaire et le délit 9 mois semble raisonnable compte tenu des nombreux points qui doivent encore faire l'objet de discussions avec les entreprises, la commission spéciale a tout de même adopté plusieurs amendements pendant à restreindre le Champ de celle-ci et à garantir l'esprit d'origine de la relation de confiance technique expérimentée en 2013, 2014 et à la satisfaction des entreprises, l'objectif est que la nouvelle relation de confiance ne se résume pas à une énième procédure de rescrit en cours d'exercice mais quel consiste bien accompagner les entreprises en amont du dépôt des comptes avec des agents issus de différents services et dans la mesure des moyens disponibles donc défavorable. Merci monsieur le ministre a allié du gouvernement. Oui, madame la présidente, l'avis est défavorable pour les arguments extrêmement proches de ceux présentés par Madame la rapporteur je saisis simplement l'occasion de cette explication, en tous cas de cet avis, pour souligner au rappeler que le gouvernement a dit être plus à l'aise avec la rédaction issue des travaux de l'Assemblée, plutôt qu'avec la rédaction, issu de la commission spéciale, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées par votre commission qui nous paraissent peut-être plus difficile à interpréter, société en malgré cette réserve, nous tenons évidemment à cet article et l'avis est défavorable à l'amendement de suppression qui est proposé. Eh bien, nous passons donc. Au vote sur l'amendement 140 avec avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Merci madame la présidente, cette habilitation par ordonnance à expérimenter l'accompagnement d'entreprises par l'administration dans la gestion de leurs obligations déclara Trives prévoit dans sa rédaction actuelle que c'est un accompagnement peut-être, je cite le cas échéant dans un cadre contractuel, la portée exacte de ce terme pose question de quelle forme de contractualisation avec une libre décision, département par département, nous le savons, cela se pratique certains agents cultive le principe de précaution, d'autres la bienveillance flou nous amène donc à demander la suppression de cette expression. Merci madame de la travée de la commission Madame Grenier. Oui, madame la présidente, ce sera un avis défavorable, cette précision est ajouté par la commission spéciale et, à l'initiative de votre rapporteur, l'une des grandes vertus de la relation de confiance, telle qu'elle a été expérimentée en 2013, 2014 était précisément son caractère contractuel, elle ne reposaient sur aucune disposition législative spécifique mais été formalisé par un protocole de coopération entre l'administration et une entreprise et résilier à tout moment, qui définissait les modalités pratiques de la revue périodicité des interventions les interlocuteurs et composition de l'équipe ainsi que les opérations examiné et qui fixait les engagements respectifs de chacune des parties, il importe de préserver c'est esprit d'origine, sauf à risquer que la relation de confiance dans sa nouvelle version ne se résume à un nouveau rescrit ou à une nouvelle forme de contrôle fiscal à la demande, la formulation retenue demeure toutefois suffisamment ouverte, le cas échéant pour laisser au dispositif, une certaine flexibilité en fonction des cires. Constance, donc avis défavorable pour la suppression de cette cette mention. Merci madame la rapporteur, Monsieur le Ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présidente, je dit il y a un instant que la nouvelle rédaction de l'article 7 ne nous paraissait pas nécessairement optimale regarde son objectif dans la mesure où celle-ci contraint excessivement le format de la future relation de confiance que l'ordonnance a vocation à définir la mention que l'amendement Madame Delattre se propose de supprimer ne ne sont pas nécessaires et source d'interrogations et même d'ambiguïté si l'expérimentation de la relation de confiance s'est traduite par la signature de conventions ces conventions ne peuvent pas bien entendu déroger aux règles sur l'acier des impôts et il va de soi que l'administration fiscale ne peut pas déroger par contrat à la loi fiscale, par conséquent, la proposition de contractualisation ne peut pas porter sur la teneur du droit applicable, il me semble que c'est une clarification qu'il est nécessaire de faire votre amendement, il participe en cohérence avec le sentiment du gouvernement sur la rédaction actuelle de l'article 7 c'est un avis favorable à l'amendement vous présente. Alors nous avons donc sur cet amendement 178 rectifié, que je mets au voire un avis défavorable de la commission. Et un avis favorable du gouvernement, donc nous allons vous procéder au vote qui est pour. Qui est con. Qui s'abstient l'amendement 178 rectifier n'est pas adopté un moment 213 présenté. Par Madame Grenier, au nom de la commission spéciale. Madame la présidente, il s'agit d'un amendement de clarification. Merci madame la rapporteure avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci, on aime la présidente, il ne semble Madame important, nous n'avons pas tout à fait la même définition de la clarification ça j'entends Monsieur le président, qui vous paraît, mais comme nous craignons depuis un petit moment et j'essaye de le dire aussi poliment possible que l'article 7 justement dans sa rédaction initiale a peut-être un peu plus de lumière justement et et que nous souhaitons et retravailler à l'occasion de la navette parlementaire, je veux simplement dire à Madame la rapporteure que si nous comprenons le sens de son amendement, nous ne pouvons pas y souscrire en l'état. Pour offrir aux entreprises un accompagnement juridique de qualité, le point clé la compétence des services et le texte adopté en commission prévoit de créer de nouvelles équipes mixtes, composées de fonctionnaires issus des services de gestion des entreprises et des services de contrôle votre amendement vise à préciser que les équipes dédiées à la sécurité juridique des entreprises serait distincte des services de contrôle et de gestion et, ce faisant, il tend à poser un principe d'organisation des services chargés d'appliquer les dispositions prévues par cet article, et donc nous ne pouvons pas être favorable au fait de fixer par la loi, un principe d'organisation des services de l'État. Merci monsieur le ministre, nous avons donc un avis défavorable du gouvernement je mais on voit l'amendement 213 qui nous a été présentée par Madame la rapporte. Sera qui est pour. C'est quoi. Qui s'abstient l'amendement 213 et adopté. Amendement 179 rectifié présenté par Madame de la. Oui, simplement pour exprimer le fait que notre surprise que certains types de d'entreprise puis théâtre puissent être privilégiée, qu'elles soient grande innovante virgule avec des enjeux fiscaux significatifs, c'est vrai que ça nous semble quelque peu approximatif sur ces enjeux par rapport à la loi qui nous est présentée. Merci, cher collègue Madame la rapporteure. Ce sera un avis défavorable lors de l'audition du directeur général des finances publiques, il nous a dit que pour que le dispositif de la relation de confiance soit ambitieux, il fallait aussi admettre qu'il ne pourra pas être ouvert à tout le monde, donc, de fait, il correspond plus naturellement aux grandes entreprises qui effectivement des sujets fiscaux importants, avec des difficultés, on a dit Ron interprétation ou aux PME qui présentent des enjeux spécifiques, notamment en matière d'innovation où effectivement les textes sont parfois pas forcément adapté parce que c'est justement une nouvelle activité, et aussi en matière de recherche, de développement et à l'international, donc ont tenu des moyens humains limités de l'administration et pour respecter le principe d'égalité devant l'impôt, il est impératif de définir ces critères de manière objective, donc un avis défavorable. Merci donc nous avons un avis défavorable de la commission de ce mini. L'avis du gouvernement. Madame la présidente, autant je rejoignais Madame Delatte sur un moment précédent autant sur celui-ci, je me rallie à la position de de la rapporteure, quelle que soit l'appréciation globale de la rédaction de l'article 7 la mention qui apparaît ainsi permis différenciés, les conditions dans lesquelles ces dispositions pour être pourront être appliqués aux entreprises, on peut considérer que leur maintien entrepris ce n'est pas la taille qui compte et que chacun doit être en capacité d'avoir les mêmes droits, en réalité, mais ces dispositions nous permettra aussi d'affiner les dispositions pourrons appliquer aux entreprises et de prévoir d'accompagner toutes les entreprises, mais avec des modalités adaptées, donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. monsieur le ministre Madame Delatte, vous maintenez votre amendement. Non, retraite. Retrait de l'amendement 179 rectifiée merci, cher collègue, nous, nous allons donc voté l'article 7 qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient, l'article 7 est adoptée après l'article 7 un amendement s'. 166 présenté par Madame La Mure. Merci madame la présidente, cet amendement reprend l'une des propositions du rapport de nos collègues Michel passe par Claude nous assure la transmission d'entreprise en France et il vise un changement de paradigme, pour faire évoluer l'administration sanction vers l'administration, conseils en s'appuyant sur une évaluation des services de l'administration, si l'offre une traduction concrète à la déclaration de principes qui figure à l'annexe de l'article 1 de ce projet de loi et qui prévoit des évaluations régulières de l'administration, associant les personnes intéressées l'amendement tend donc à instaurer une évaluation appelé à porter non seulement sur les services locaux de l'administration fiscale, mais également sur les services des autres administrations dont l'action peut avoir un impact sur la vie des entreprises. Merci madame Lamure avis de la commission Madame Grenier. Merci madame la présidente, n'est pas possible de contraindre par la loi le 1er ministre a entamé une telle démarche, il aurait fallu que la loi fixe un cadre aux évaluations prévues et que, en application de ces dispositions, le 1er ministre prenne des décrets d'application, mais ce n'est pas ce que prévoit cet amendement et donc je ne peux pas il y a trop favorable donc demande de retrait. Ou, à défaut, avis défavorable, je suis désolé madame Lamure. Merci madame la rapporteure, allié du gouvernement Monsieur miné. Merci madame la présidente, je ne peut que compatir avec la peine de madame Lamure Lamure cet amendement, puisque depuis quelques heures maintenant, j'ai subi les mêmes avis défavorable de Madame la rapporteur à une différence près: c'est qu'elle ne va pas encore dit qu'elle était désolée mais je ne désespère pas et peut-être que la soirée ne permettra de diarrhée plus sérieusement la l'idée ouvertement et défavorable à l'amendement que vous portez pour pour les mêmes raisons compris sur les conditions d'appréciation et par le fait que la stratégie nationale de l'action publique définie au début de ce projet renvoie un horizon 2020, 2 qui ne permettrait pas de de mettre en 9 l'amendement que vous nous proposez donc éviter favorable, demandes de retrait. Merci monsieur le ministre madame Lamure. Oui, voilà encore, je comprends que, peut-être, sur le fond, vous seriez d'accord mais que c'est une question de de forme, ou une question technique, donc avec regret, j'accepte le retirer. Merci, cher collègue, l'amendement 166 et donc retiré article 7 bis, un amendement 180 rectifié présenté par Madame de la. Oui, madame la présidente, cet article, introduit en commission spéciale et qui modulent l'annulation d'exonération de cotisations sociales en cas de travail partiellement dissimulé n'entre pas pour nous dans le Champ du droit à l'erreur, puisqu'il se fait généralement en connaissance de cause, la non-déclaration de salariés par leur employeur et plus souvent le fruit d'une tentative de fraude que d'un oubli ou d'une erreur, alors au vu des conséquences financières et sociales néfaste pour le salarié, les proposé de supprimer cet article. Oui merci madame la présidente, alors cet article additionnel provient de nos échanges au cours des auditions avec Lacoste, qui chapeaute le réseau des Urssaf constat de de dans le contrat de travail dissimulé dresser l'employeur perd le bénéfice des exonérations de cotisations sociales dont il a bénéficié s'ajoutent au redressement assorti de majorations et, le cas échéant à des poursuites pénales cette peine complémentaire correspond à la volonté de lutter efficacement contre le travail dissimulé, toutefois, la notion de travail dissimulé, recouvre des situations assez différentes les unes des autres, il peut s'agir bien annonce tendue devrait fraude mais également d'un oubli portant sur quelques heures supplémentaires ou encore de la requalification en travail salarié d'une prestation de travail indépendant, on peut s'interroger sur la pertinence de punir avec la même sévérité ces manquements de nature différente et surtout l'annulation totale des exonérations dont l'employeur a pu bénéficier peut apparaître excessive dans les cas où le montant des rémunérations que l'Urssaf considère comme dissimulé est dérisoire par rapport au montant dans l'entreprise s'est régulièrement acquittée, cette situation a tendance a renforcé la méfiance des employeurs vis-à-vis des contrôles des Urssaf alors l'article 7 bis visant que l'ampleur de la sanction complémentaire soit plus en rapport avec l'ampleur de la dissimulation, résulte donc de nos échanges avec la cause s'agit bien entendu de ne pas préserver je dirais privilégié. Les fraudes éventuelles à l'administration mais c'est vraiment je sûr qu'il y a des des où effectivement de bonne foi et des heures supplémentaires qu'on pas été déclarés, mais dans un nombre moindre et quant à la requalification travail salarié d'une prestation de travail indépendant, moi je peux vous dire qu'il y a souvent souvent les personnes qui ne qui ne qui méconnaissent, en fait, cette disposition et qui se trouve effectivement dans une situation par rapport à l'Urssaf frauduleuses alors qu'ils le font en toute bonne foi, franchement sur sur cet amendement et moi j'en, j'entends bien ce que ce que vous mais on a vraiment voulu bien bien bordé pour effectivement que ce soit pas la porte ouverte aux fraudes donc un avis défavorable sur l'amendement. Merci madame la rapporteur, Monsieur le Ministre à vie du gouvernement. Merci, on a la présidente le gouvernement partage l'avis de Madame Delattre, la proposition d'amendement qui est porté, nous considérons comme vous, Madame la sénatrice, que dans le cas traités par cet article, l'essentiel des faits constatés relèvent d'une tentative de fraude ou dissimulation, il nous considérons par ailleurs que dans la mesure où depuis le début du débat sur le droit à l'erreur, nous disons, nous répétons que ce droit à l'erreur ne s'applique pas lorsqu'il y a une volonté frauduleuse, ça serait envoyer un signal incohérent contreproductif que de maintenir une telle disposition dans le texte, pour laquelle le gouvernement souhaite que cet article soit supprimé soutient l'amendement déposé par Madame De Lattre. Merci monsieur le ministre, nous allons mettre au voile amendement 180 rectifier avec un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement qui est pour.

Qui s'abstient, l'article 7 bis est adopté article 8, une demande de paroles de Madame Françoise Ferrat. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, les objectifs du projet de loi état au service d'une société de confiance entend enclencher une dynamique de transformation de l'action publique en renforçant le cadre d'une relation de confiance entre le public et l'administration, pour ce faire, il pose d'une part les jalons de cette relation accompagnement engagement et dialogue et d'autre part, il vise à rendre l'action publique plus efficace, plus moderne et plus 5 l'ensemble des députés ont compris ce texte, en effet, ils ont introduit à l'Assemblée nationale à l'article 8 qui suit un alinéa, mettre en place une véritable mesure de simplification administrative, répondant aux objectifs du présent projet de loi cette mesure très attendue par les filières agricoles et juste quoi qui recourent de manière importante au contrat saisonnier, notamment lors de la récolte permet l'émission d'un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d'un saisonnier est inférieure à un mois mais à cheval sur 2 mois distincts, je prendrai l'exemple des vendanges en Champagne si vous débutez vendanges le 31 août pour les poursuivre les premiers jours de septembre vous étiez tenue jusqu'aujourd'hui, a préparé 2 fiches de salaire, cet amendement est une réelle simplification ainsi avec quelques-uns de mes collègues nous avions déposé un amendement complétant cette disposition nouvelle dans le droit actuel, le code rural et celui de la Sécurité sociale, définit la rémunération prise en compte pour la réduction des charges patronales accordée pour l'embauche demandeurs occasionnels, or dans ce cas, le calcul ne se fait pas sur la totalité du contrat de travail maintenant chaque mois civil ainsi en complément d'une mesure validés à l'Assemblée nationale, notre amendement visait à prendre en compte la durée totale de travail du contrat saisonnier sans effet couperet à la fin d'un mois civil. Seulement de travaux non n'a pas été retenu au titre du fameux article 45 de la Constitution, au motif qu'il n'aurait pas de lien, même indirect avec le texte, excusez moi, ça me semble un petit peu absurde et à l'heure où nous prenons la simplification, c'est bien dommage, je vous remercie, Monsieur le Ministre de prendre en compte cette mesure de complément de simplification que manifestement le Sénat ne semble pas légitime à porter.

relatives au contrôle de l'application du droit du travail ouvre la possibilité pour la directe de prononcer des amendes administratives en cas de manquement à certaines dispositions du droit du travail, l'article 8, propose, lui, que ces amendes puisse être remplacée par un simple avertissement, il serait donc possible pour les agents de la Directs de choisir l'avertissement plutôt que l'amende administrative en cas de manquement au droit du travail, mais rappelons-nous ici de quels manquements nous parlons, durée maximale du travail, respect du repos quotidien, salaire minimum respect des obligations des employeurs en matière d'installations sanitaires, de restauration et d'hébergement loin de considérer que ces manquements sont bénins, les agents de contrôle. Font déjà grandement usage du rappel à la loi plutôt qu'à l'amende sur 160400 sur 160469 pardon d'observation rédigé par des agents du contrôle, seuls 429 décisions ont abouti à une amende et qu'en l'état actuel du droit, il est déjà permis à l'employeur de contester la décision des contrôleurs au tribunal et ministre et qu'en cas d'amende le contrôleur doit prendre en compte des circonstances et la gravité du manquement du comportement de son auteur et de ses ressources et ses charges, cela est tellement vrai que le rapport du Sénat lui-même nous dit, je cite, que l'on peut donc considérer qu'il existe déjà en la matière, une forme de droit à l'erreur pour l'employeur qui est laissée à l'appréciation des agents de l'inspection du travail et que par conséquent, cet article ne s'appliquera que dans les cas rare en pratique dans lesquels un agent de contrôle considérait qu'un manquement est suffisamment grave pour justifier la transmission d'un rapport, mais où la Direct et estimerait qu'une sanction pécuniaire n'est pas justifiée ajouté que les contrôleurs doivent prendre en compte la bonne foi de l'employeur paraît redondant avec l'article L 95 IV qui prévoit que pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte des circonstances et la gravité du manquement le comportement de son auteur, ainsi que ses ressources et ses charges, enfin les contrôles et la sanction des fraudes sont inhérents échos relatifs au système déclaratif et au respect de l'ordre public, économique et sociale, autant de raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article. Merci, Monsieur, Madame Bruni-avait de la commission. Merci madame la présidente, que le manquement qu'il a constaté justifie qu'qui transmettent un rapport au Direct ce dernier prononce en général une amende administrative les avertissements ne seront prononcées que dans les cas qui sont rares en pratique dans lesquelles le directe, juge qu'il n'est pas opportun de prononcer une amende mais souhaite néanmoins rappeler formellement l'employeur à ses obligations, dans ces cas, il peut être pertinent prononcer un avertissement plutôt que de classer sans suite une saisine de l'inspection du travail, donc la commission spéciale a émis un avis défavorable à cet amendement de suppression. Merci madame la rapporteure à vie du gouvernement Monsieur miné. Merci madame la présidente, la vie est défavorable, aussi, j'ai eu l'occasion de dire lors de l'intervention en discussion j'en discussion générale que c'était pour nous une mesure emblématique et que si l'administration et notamment l'inspection du travail était en capacité délivre un carton rouge, fait aussi savoir délivre un carton jaune pour reprendre une expression ou une image nous considérons véritablement qu'il y a lieu de créer ce dispositif pour qu'un certain nombre d'entreprises puissent être rappelés à leurs obligations, mais en considérant que, du fait de leur bonne foi, du fait de la faible importance des faits constatés cette sanction par avertissement serait suffisante, sans qu'il y a lieu de fixer une amende, donc l'avis défavorable. Merci monsieur le ministre, explications de vote de Madame Tallien pollueurs,

de l'inspection du travail ou par leur hiérarchie et que donc cette mesure dite emblématique étant faite à toute communication beaucoup de communication, mais sans réel impact parce que l'inspection du travail ne ne ne va pas directement à à l'amende pourcent qu'il n'y aura pas forcément énormément de, de, d'évolution en réalité avec cet article, par contre, là où nous attirons l'attention, et là ce serait peut-être une mesure emblématique d'un une volonté du gouvernement qui démontrerait la volonté du gouvernement effectivement de, de, de véritablement mettre des moyens pour faire en sorte que le droit du travail, ce qu'il en reste soit respecté, ce serait de recommencer à embaucher des inspecteurs du travail, car le nombre des agents de contrôle de l'inspection du travail a énormément baissé, et dans le le projet de loi de finances 2017 une nouvelle baisse a été enregistrée, on a beaucoup moins de postes mis au concours que de départ à la retraite et ce qu'on observe sur le terrain, c'est, c'est peut-être de de donner un peu un carton rouge au gouvernement là-dessus, hein, on veut faire de la communication en disant qu'on sera plus souple, on est surtout plus souple casse parce qu'on est moins présent sur le terrain et je pense que ce n'est pas un bon signal envoyé à ceux qui souhaitent, je dirais, être un petit peu libre vis-à-vis du code du travail qui est déjà bien alléger. Merci, cher collègue. Nous allons mettre au voile l'amendement 141 ans, qui a un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est court. Qui s'abstient l'amendement 141 n'est pas adopté, amendement 177 présentée par Madame Lamure. Oui, madame la présidente, introduite par un amendement du groupe Nouvelle Gauche, à l'Assemblée nationale, pour lequel le gouvernement s'en était remis à la sagesse des députés, cette disposition propose un alourdissement de la sanction existante en cas de réitération du manquement après un avertissement procédure que le projet de loi crée par ailleurs, le montant de l'amende serait majorée de 50 pourcent lorsque l'employeur a déjà reçu un avertissement au cours de l'année écoulée en cas de récidive dans un délai d'un an, le plafond de l'amende administrative qui peut être prononcée par la directe serait doublé la commission spéciale du Sénat a proposé de préciser que ces majorations ne serait applicable qu'en cas de nouveaux manquements de même nature, toutefois ce message de fermeté particulier adressé aux entreprises brouille le message général de bienveillance instituant un droit à l'erreur, cet amendement vise donc à supprimer cette disposition, ce qui donnerait le signal de la cohérence de la parole publique en direction des entreprises. Merci, cher collègue, avis de la commission Madame le rapporteur. Oui merci madame la présidente, alors contrairement à ce que semble indiquer l'objet de l'amendement les dispositions qu'il vise à supprimer, ne prévoit pas une majoration du montant de l'amende, mais une majoration de son montant maximal il revient en Direct de moduler ce montant en fonction des circonstances alors je précise que le montant moyen des amendes prononcées est aujourd'hui proche de 500 euros soit nettement en deçà du plafond de 2000 euros par salarié concerné, en outre, la majoration du montant de l'amende en cas de récidive semble nécessaire pour que l'avertissement est réellement une valeur préventive et enfin la proposition d'amendement revient sur une présient Sion qui, précision qui a été adopté par la commission spéciale et qui me semble utile, à savoir que la majoration des plafonds d'amende en cas de récidive s'applique dans le cas d'un nouveau manquement de même nature que le 1er donc pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable à cet amendement.

il est normal qu'en cas de récidive sur des faits de même nature, la sanction puisse être considérée comme pouvant être plus grave puisque l'information : l'avertissement a été fait et donc, en cohérence avec la position tenue à l'Assemblée nationale et et en partageant les amendes, les arguments pardon évoqués par Madame la rapporteur d'avis défavorable. Merci monsieur le ministre, nous allons à madame Lamure. Explique oui mais la présidente simplement contenu que la commission spéciale en quelque sorte adouci le le l'amende, moi je suis d'accord pour retirer cet amendement. Eh bien, merci, cher collègue. L'amendement 167 retiré, nous passons à l'amendement 104 qui est présenté par Madame Paul y en. Merci madame la présidente, nous souhaitons participer à lutter contre la fraude et travail illégal, notamment par des propositions et notamment sur l'efficacité des services d'inspection du travail et notamment pour proposer pourront plus efficient, les dispositifs d'investigation des pouvoirs publics en la matière, guidé par la rationalisation de l'action de l'État et par le renforcement de l'aide de l'efficacité de la réponse pénale vis-à-vis de la délinquance sociale nous demandons, nous proposons que soit menée une réflexion sur l'opportunité de la création d'un service de l'inspection judiciaire du travail, alors nous aurions pu déposer un amendement qui crée ce service mais nous, nous, un petit peu la crainte que l'article 40 nous soit appliqué, il faut dire que lors de l'examen de ce projet de loi différents articles dit recevabilité ont été largement appliqué, donc, malgré le fait qu'on sait que nous savons que les rapports ne sont pas très appréciés dans cet hémicycle, nous avons préféré donc vous proposer cela par une demande de rapport 2 exemples viennent appuyer la pertinence de mener cette réflexion, le 1er est la création du service de douane judiciaire créée lorsque la lutte contre la contrefaçon est devenu une priorité de l'action publique, le second est d'actualité et l'annonce récente par le gouvernement de la création d'un service d'enquête judiciaire sur les affaires de fraude fiscale, disposant d'une compétence nationale et opérationnel d'ici à 18 mois, en parallèle, nous proposons donc la création d'un service de l'inspection judiciaire du travail, en effet, pour mener à bien ses missions, l'inspection du travail, dispose d'un certain nombre de prérogatives néanmoins certaines situations, notamment les plus complexes, tels que les enquêtes suite à un accident grave ou mortel, les contrôles coordonnés en matière de lutte contre le travail illégal ou les fraudes au détachement la traite contre les êtres humains etc nécessite souvent lorsque l'inspection du travail est à l'initiative d'une procédure pénale des investigations complémentaires de la part d'un service de police judiciaire, or ces interventions sont à l'allonge la durée de traitement des procédures, les actes d'investigation sont redondants et parfois les mis en cause ont ont disparu entre la découverte de l'infraction et la possibilité, tenue d'un procès verbal donc afin de résorber ces difficultés, il pourrait être créer un service dépendant du ministère du Travail, qui se composerait d'inspecteurs et de contrôleurs du travail investie des prérogatives de police judiciaire sur le Champ du droit pénal du travail dans un schéma organisationnel, proche de celui des douanes judiciaires voilà, nous comptons sur votre écoutez votre réponse Monsieur le ministre pour prendre en considération cette proposition qui vise véritablement à renforcer l'efficacité des services de l'inspection du travail. Merci, cher collègue, Madame Bruni-avis de la commission. commission. La présidente, ce sera un avis défavorable, déjà conformément à la position désormais traditionnel du Sénat, la commission spéciale a émis un favorable à cette demande de rapport, je note par ailleurs que l'objet de l'amendement est relativement long et détaillé et que l'on pourrait presque considérer que les auteurs de l'amendement déjà rédigé le rapport qu'il demande au gouvernement ainsi soit le gouvernement est favorable à la création d'service d'inspection judiciaire du travail et il lui appartient alors de soumettre au Parlement un projet en ce sens en swahili est défavorable et le rapport qu'il remettra au Parlement serait nécessairement décevant pour les auteurs de l'amendement, donc avis défavorable. Merci madame la rapporteur, Monsieur le Ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présidente, pour dire d'abord que, à titre personnel et peut-être vont être les les 10 passe à l'Assemblée, je partage la position du Sénat sur l'inopportunité des rapports de monde gouvernement puisque souvent d'ailleurs ils ne sont pas nécessairement rédigé et quand ils sont rédigés ne sont pas nécessairement donc je considère, je considère Madame la sénatrice, mesdames et messieurs les sénateurs, que le plus souvent les plus efficaces, ce sont, c'est que les parlementaires se saisissent de leurs prérogatives en terme de mission d'information de commission d'enquête quand c'est nécessaire pour mener ce travail au-delà de cette position de principe sur les rapports le dispositif que vous proposez d'étudier dans le le rapport que vous souhaitez du gouvernement se heurte à 2 difficultés qui nous amène à donner un avis défavorable. D'une part la création d'inspection du travail judiciaire, placée sous l'autorité des parkings mais connaîtrait des dispositions de l'article 4 de la convention numéro 91 qui place, inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale unique principe que le présent projet de loi renforce dans l'introduction du nouvel article L. 80 21 tirez un dans le code du travail, ce principe a été rappelé dans un récent avis du Conseil national de l'instruction du travail qui dit que, si la convention numéro 81 n'impose pas, en elle-même un modèle d'organisation et laisse aux autorités nationales, une possibilité d'adaptation de l'organisation du système d'inspection en considération des conditions de leur exercice elle exige qu'une autorité centrale soit chargée d'assurer la surveillance et le contrôle des inspecteurs dans des conditions propres à garantir leur indépendance et le respect des dispositions de cette convention, et par ailleurs la proposition que vous formulez connaît également les dispositions de l'article 17 de la même convention relative à la liberté de suite que les inspecteurs du travail peuvent donner leur contrôle puisque c'est suite serait nécessairement judiciaire et donc cela me connaître et c'est ce principe de liberté de suite enfin, il convient de rappeler que le lien de confiance entre l'inspection du travail des entreprises s'appuie sur le fait que les inspecteurs du travail, assure un suivi global des entreprises et une connaissance et aux connaissances pardon lorsqu'il donne des suites à leur contrôle du contexte social et économique de l'entreprise, contexte qui tiennent largement compte pour notifier de manière privilégiée d'observations et non des sanctions et la création d'un service judiciaire d'inspection du travail, en privilégiant une approche non pas l'entreprise Montparnasse. Claude nous paraît plutôt de nature à rompre ce lien en tout cas, porte le risque mais principalement pour les 2 articles de la convention de l'OIT qui serait méconnu par la proposition, vous portez, nous ne pouvons donner suite favorable à votre demande, Rabat. Merci monsieur le ministre a, je vais donc mettre à explications de vote, chers collègues. Oui, alors je je trouve dommage que la commission s'exprime uniquement finalement sur sur la sur la forme par rapport à, à ce que vous m'avez répondu monsieur mise, bon je sur l'Organisation internationale du travail je vais regarder ça ça de près, mais sur la liberté de suites judiciaires, je comprends pas très bien lorsqu'un inspecteur du travail, dresse un procès-verbal, il transmet bien tout cela, un juge qui prend la main après donc je je comprends pas, et là ce serait aussi la constitution de ce dossier qui permettraient d'aller bien plus vite parce que les inspecteurs du travail aurait d'ores et déjà des prérogatives de police judiciaire et ça permettrait une meilleure efficacité de de ces procédures, donc j'avoue ne pas bien comprendre je je je reviendrai certainement dans le cadre notamment peut-être une proposition de loi sur sur cette sur je pense de véritablement de nature à à rendre plus efficace, les services de l'inspection du travail et non pas de rompre le lien car il s'agirait d'un service, je dirais, à part les justement qui permettrait aux inspecteurs du travail de, de, de, de tout de suite de passer le relais sur des des affaires véritablement avec des objets très lourd et de se consacrer pleinement à leur à leur mission plus de terrain, voilà, donc je pense que là il y a peut-être une une légère incompréhension sur ce que ça pourrait donner sur le terrain, je vous remercie. Madame Sophie Calle polluant dit qu'il n'y a pas de réponse sur le fond, donc moi je vais lui donner une réponse sur le fond et pas sur la forme de de ma part, je ne suis pas la commission, je crois qu'il y a une erreur ou un vrai contresens sur le rôle de l'inspection du travail dans cet amendement, l'inspecteur du travail, c'est celui qui veille à l'application du droit dans l'entreprise, mais c'est aussi sans doute surtout celui qui assiste le chef d'entreprise dans l'application de ce droit du travail et qui a donc un rôle selon le code du travail de conseil des chefs d'entreprise, ce qui me gêne profondément dans l'amendement qui est proposé, c'est qu'on ne fait plus de l'inspecteur du travail, un partenaire de l'entreprise quelqu'un qui est dans le lien de confiance avec le chef d'entreprise, mais bien d'un policier c'est c'est-à-dire qui est qu'un qui va inspecter et on sait déjà que chez les chefs d'entreprise, c'est déjà trop souvent vécu comme cela, l'inspecteur du travail a déjà trop souvent vécu comme quelqu'un qui s'immisce de façon intrusive et de façon policière dans l'entreprise, donc il y a, à mon sens d'abord une erreur sur le fond, sur le rôle de l'inspection du travail et ensuite un mauvais une mauvaise manière faite aux inspecteurs du travail, parce que ça n'est pas leur rendre service que de les placer dans un rôle de police judiciaire qui n'est pas du tout leur rôle après d'expérience, je peux vous dire que, en cas d'accident grave c'est ça surtout qui est lié, qui est visé, il y a effectivement 2 enquêtes, une enquête de de l'inspection du travail, une enquête des services de police judiciaire qui travaillent main dans la main qui sont complémentaires, vraiment, je crois qu'il ne faut pas, il faut faire très attention à ne pas mélanger les 2 genres et re-c'est le rôle de l'inspecteur du travail qui est celui de conseiller d'entreprise, vous aurez compris que je ne suis pas favorable, c'est un moment. Merci, cher collègue, s'il n'y a plus de demande, explications de vote. Je vais mettre au voile amendement 104 qui a un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est. Qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté, je maison voilà Rettig le 8 qui est pour.

et un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune un amendement 45 présenté par le gouvernement. Merci madame la présidente, l'article 10 du projet de loi initial introduit une disposition et ont pour objet de permettent l'extension du mécanisme de rescrit ils venaient ainsi compléter des dispositifs relativement anciens, comme le rescrit en matière fiscale ou plus récents tels que les risques sur l'ordonnance du 10 décembre 2015, l'article 10 renvoyé dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale : un décret le soin de préciser le Champ d'application de cette extension votre commission a supprimé cet article au motif de son inconstitutionnalité en se fondant sur l'avis du Conseil d'État en ne précisant pas les domaines le législateur ferait selon vous, Oeuvres d'incompétence négative vous répond à ces critiques, le présent amendement propose de ne plus opérer un renvoi un décret mais de procès d'emblée à l'extension envisagée, il prévoit ainsi d'être le Champ du rescrit créances identifiés par le Conseil d'État dans son étude de 2014 intitulé le rescrit sécuriser les initiatives, les projets, c'est-à-dire du rescrit qui prémunit sont bénéficiaires d'une action administrative ex-Post qui aurait pour effet de mettre à sa charge une somme d'argent suivant notamment les préconisations du Conseil d'État le présent amendement développe 5 nouveaux dispositifs de rescrit affaire afférents à la fiscalité de l'aménagement à la taxe perçue par la région Île-de-France en application des articles L. 100 120 tirer 1 et suivants du Code de l'urbanisme redevances des agences de l'eau et à la redevance de l'archéologie préventive.

et ensuite on verra d'abord le sous-hommes d'abord le sous-amendement que vous présentez. Bien le sous-amendement que je vous propose, apporte un certain nombre de précisions, prenant l'exemple des dispositions existantes en matière de rescrit ainsi que sur la première version de l'article 10 du projet de loi dont vous ne de nous parler, Monsieur le Ministre, cet amendement, qui a précisé que les réponses apportées sont opposables par le demandeur à l'administration, jusqu'à ce qu'elle intervienne un chargement de fait ou de droit,

Ce qui concerne l'amendement que vous avez déposé Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé cet amendement vise à réintroduire l'article 10 que nous avons supprimé en commission Alain modifiant sensiblement le contenu, l'article 10 du projet examiné en commission prévoyait d'inscrire la généralisation du recours aux rescrit Hossein du Corps de des relations entre le public et l'administration cet article y toutefois des décrets le soin de définir ses modalités, mais également son Champ d'application, nous avons donc estimé que ces dispositions étaient entachées d'incompétence négative et les avons écarté, nous nous sommes également interrogé dans notre rapport sur la pertinence de créer un régime général a matière de rescrit alors que toutes les procédures existantes existantes sont très spécifiques et sont prévues: d'année texte sectorielles, le gouvernement semble avoir tenu compte de nos remarques puisque la réécriture qui proposent de l'article 10 introduit rescrit spécifique dans 5 secteurs et que ces dispositions doivent directement c'est serré dans les codes concernés, à savoir le code de l'urbanisme pour la taxe d'aménagement, le versement pour soudain cité et la taxe pour la construction de certains locaux en Île de France, le corps de l'environnement pour les agences de l'eau et en fait, le code du Patrimoine a matière de redevances d'archéologie préventive j'aime donc un avis favorable à l'adoption de cet amendement, sous réserve de l'adoption de sous amendements que je vous ai présenté il y a quelques secondes, prenant l'exemple des dispositions existantes en matière de rescrit ainsi que sur la première version de l'article 10 ce sous-amendement de temps, a précisé que les réponses apportées sont opposables jusqu'à ce qu'elle intervienne un chargement de fait ou de droit, aucune nouvelle position soit notifiée au demandeur, donc un avis favorable. Merci Monsieur Lüscher Monsieur le Ministre quel Avedon, le gouvernement sur le sous-amendement. Madame la présidente, d'abord pour dire à monsieur le rapporteur qui, effectivement, le gouvernement a tenu compte des observations et de la position tenue par la commission spéciale au sujet de l'article dit : dans sa rédaction initiale, d'où la présentation ce soir devant vous, d'un amendement différemment rédigé et répondant à ces observations, pour ce qui concerne le sous-amendement, vous nous proposez, les précisions qui sont apportées sont des précisions utiles qui facilite aussi l'intelligibilité du dispositif que nous proposons donc, la vie est favorable sous-amendements en souhaitant et en félicitant peut-être par avance qu'il permette l'adoption de l'article de Merci monsieur le ministre je commence donc par mettre aux voix l'amendement 214 qui était présenté par Monsieur Lucho au nom de la commission spéciale qu'il y a donc un avis favorable du gouvernement qui est pour.

Alors, à l'article 11 qui est supprimé, nous avons un amendement 46 présenté par le gouvernement Monsieur miné. Oui, madame la présidente, dès lors que le gouvernement dans son amendement numéro 45 que vous venez d'adopter propose adopter des dispositions créant de nouvelles formes de réinscrire l'article 10, nous vous proposons corrélativement, de rétablir l'article 11 qui permet d'expérimenter pour certains des risques ainsi créer un dispositif de silence vaut accord à l'issue d'un délai de 3 ans, lorsque le demandeur présente un projet de prise de position formelle, une démarche de silence vaut accord dans le domaine du rescrit constitue pour nous un pas supplémentaire dans l'institution d'une relation de confiance entre usagers, administration, celle-ci ne répond pas, un projet de rescrit elle est réputée l'approuver et l'expérimenté en matière de Paris essentiel, c'est le sens de cet amendement de rétablissement de l'article. Merci monsieur le ministre, un avis de la Commission, monsieur L'article 11 a été supprimé en commission par cohérence avec la suppression de l'article 10 se fondant sur cette dispositions il prévoyait la mise en place à titre expérimental de mécanismes permettant à l'administration d'accepter tacitement une proposition de rescrit 13 mise par un usager, l'amendement du gouvernement vise ici à réintroduire ce mécanisme expérimental sur la base donne décrit dans les secteurs concernés par des procédures réintroduites à l'article 10 je m'interroge sur cette procédure chez les services concernés devront déjà se familiariser avec les nouvelles procédures prévues à l'article 10 il risque donc d'éprouver certaines difficultés pour appliquer ce nouveau dispositif expérimental en même temps des erreurs matérielles de traitement pourrait à l'autre, avoir des conséquences très dommageable à cause du principe même de l'acceptation tacite, je pense donc qu'il est prématuré ou trop tôt pour mettre en oeuvre cette procédure expérimentale et de ce fait une demande de retrait ou un avis défavorable. le je, je vais donc mettre aux voix l'amendement 46 qui fait l'objet d'un avis défavorable ou d'un retrait, monsieur le ministre, nous maintenons donc cet amendement aux voix donc, qui est pour. Quoi. Qui s'abstient l'amendement 46 n'est pas adoptée et l'article 11 reste donc supprimé après l'Artic. Le 11 nous avons un amendement 58 présenté par le gouvernement Monsieur le ministre. Merci madame la présidente, avant de devenir le le droit commun, la règle du silence vaut acceptation pouvaient être instituée ponctuellement par voie réglementaire, mais institution du principe du principe du silence vaut acceptation par la loi du 12 novembre 2013 a conduit le législateur à prévoir des exceptions, notamment les relations entre l'administration pardon et ses agents, le principe est donc le silence vaut rejet dans les relations entre l'administration et ses propres agents, on ne peut déroger que par la loi, ce dispositif plus contraignant que le dispositif antérieur qui permettait de déroger à la règle par voie réglementaire les Suisses sont critiquables dans lesquels la simple reconduction d'une disposition réglementaire de vaut accord oblige à passer par la loi pour résoudre cette difficulté relevée par le Conseil d'État le présent amendement permet déroger par voie réglementaire, au principe du silence vaut rejet dans la dans les relations entre l'administration et ses propres agents. Merci monsieur le ministre, monsieur Buchet, avis de la commission. Cet amendement est est important gagner car il concerne la mise en oeuvre du principe selon lequel le un seul administration vaut acceptation, bien sûr, tout le monde est favorable à ce principe car il permet de simplifier les relations entre l'administration et le public, toutefois depuis 2013, son application est d'une complexité extrême en 2015 non collègue Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli ont démontré qu'il y avait davantage d'exception que l'application de la règle de fait, les citoyens sont perdus et devrait consulter 42 décrets d'application pour savoir si oui ou non, le Style, un seul administration vaut acceptation ou Roger, je répète 42 décrets une exception actuelle ce principe au moins le SIDA un s'est gardé par l'administration de un de ses relations avec ses agents vaut refus par cet amendement, le gouvernement propose de créer des exceptions à cette exception le silence gardé par l'administration de la ses relations avec ses agents vaudrait acceptation d'un certificat et rejet dans d'autres, cette situation deviendrait ubuesque, voire kafkaïenne pour nos petites communes qui sont déjà bien me peine de gérer tout à la complexité du droit de la fonction publique et qui se sentent souvent abandonnés par les préfectures, je vous ai proposé donc un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, nous allons donc mettre aux voix l'amendement 58 du gouvernement qui a un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est quoi. Qui s'abstient l'amendement 58 n'est pas adopté après l'article 11 un amendement de rectifier, présenté par Madame d'idées. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, dans son projet de loi présenté en conseil des ministres, le gouvernement avait décidé de précéder l'inscription dans la loi de la Suède jurisprudence d'Anthony cette jurisprudence du Conseil d'État établissait que tout vices de procédure dans l'élaboration d'une décision administrative l'étaient pas de nature à entraîner son annulation pour connaître d'administratif soit annulée pour vice de procédure, 2 situations sont posées la personne intéressée par là doit avoir été privés d'une garantie prévu par la procédure viciée ou le vice doit avoir exercé une influence sur le sens de la décision résultant de la procédure, dans d'autres d'Antony dans la loi permet de donner à cette règle jurisprudentielle opportune une place durable et une sacralité évidente, elle assure ainsi pleinement aux collectivités publiques qu'un vice mineur affectant la procédure d'élaboration de leurs décisions ne puisse les remettre en cause devant le juge, il s'agissait aussi d'instiller davantage de stabilité et donc de confiance dans l'activité des collectivités publiques.

Cet amendement propose de codifier la jurisprudence dite d'Anthony, du Conseil d'État, pour mémoire, selon cette jurisprudence vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalables l'entache d'illégalité, l'actuel ministre hâtif à une question que d'un ou ou 2 hypothèses : la première, Cécile a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise la 2ème si a privé les intéressés d'une garantie lors de l'examen du projet de loi par la commission spéciale, nous avons approuvé l'abrogation d'une disposition législative de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit qui était dépourvu de portée juridique depuis cette jurisprudence la commission spéciale n'a pas souhaité codifier cette même jurisprudence de dans la loi, souscrivant à l'analyse du Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi selon laquelle ce choix serait inopportun, car un trio mais il priverait le juge administratif de la possibilité de lui apporter des amendements nécessaires et afin de prendre en compte la spécificité de certaines procédures préalables sectorielles, il vous est proposé un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur et nous passons à l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, comme vient de le dire, monsieur le rapporteur, l'article 27 du projet de loi examiné dans le cadre de la procédure législation commission abroger l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 afin de tirer les conséquences des principes dégagés par la jurisprudence d'Anthony, du Conseil d'État, en date du 23 décembre 2011, en cohérence avec l'analyse du Conseil d'État lors de l'examen du projet de loi, le gouvernement estime, comme la commission n'est pas nécessaire ni opportun d'aller au-delà de cette clarification du droit applicable en consacrant par la loi d'application de la jurisprudence d'Anthony, pour nous, l'appréciation des conséquences comporte un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalables relève avant tout de l'office du juge et lequel nous paraît défini manière satisfaisante par la jurisprudence administrative et donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable.

monsieur le ministre, mais, chers collègues, je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi, afin de poursuivre l'examen de ce texte. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé, nous allons donc continuer encore pendant 30 minutes et nous allons passer à l'article 12 heures avec un amendement 142 présenté par Madame pruneaux. Merci madame la présidente, nous demandons la la suppression de de cet article en effet le problème du certificat d'information qu'il donne une vertu législative à ceux qui procèdent quasiment du simple document d'information administrative en et que c'est les attendus sont largement couverts, s'agissant des entreprises par la partie réglementaire du Code du commerce, portant notamment sur les cendres de formalités existant dans les chambres consulaires, l'avis du Conseil d'État et d'ailleurs négatif sur cet article qui n'apporte rien à l'existant et qui fait peser une nouvelle responsabilité sur l'administration d'une part et empiète sur les compétences d'autres instances, d'autre part, je cite : le Conseil d'État souligne l'intérêt que peuvent présenter des mesures tendant ta ouvrir à toute personne le droit d'obtenir de l'administration, une information exhaustive sur les normes régissant son activité économique ou sociale, il constate cependant que le projet de loi ne permet pas de résoudre à cet objectif dès lors qu'il n'est pas dans l'intention du gouvernement de prévoir que le certificat mentionne les règles relevant de chacune des administrations responsables qu'il s'agisse de l'État, des collectivités territoriales ou toute autre personne publique en matière de responsabilité de la puissance publique, le projet ne modifie pas l'état du droit qui prévoit déjà qu'elle peut être engagée en cas d'information et Renée ou incomplètes, ayant créé un dommage, en conséquence, le Conseil d'État ne retient pas cette disposition, qu'il n'estime pas nécessaire, il considère que l'objectif recherché d'accessibilité de la norme, comme le développement dans les différentes administrations de la mission d'information sur les normes auxquelles il ce cri pleinement peuvent être atteints sans création de nouvelles règles, mais par l'action de ces administrations et par conséquent par la voie de circulaires, je vous remercie. Merci, cher collègue, avis de la Commission, monsieur Luce. Cet amendement entend supprimer le certificat d'information type, je cite, que ce dispositif n'apporte rien à l'existant et qui fait peser une nouvelle responsabilité sur l'administration d'une part et empiète sur les compétences d'autres instances, d'autre part, comme les auteurs de l'amendement j'ai lu avec intérêt l'avis du Conseil d'État qui considérait en substance comme tels dispositifs n'apportait pas de plus-Value réelle par rapport aux outils d'information existants en raison en particulier de son manque d'exhaustivité, puisque chaque administration ne répondraient que sur les normes qu'la mission d'appliquer et également aussi de l'absence d'effet de cristallisation sur les règles présentées hors des auteurs de l'amendement oublie de préciser que depuis le texte initial, ces 2 écueils auront au moins en partie étaient traités, à défaut de pouvoir créer des à présent un guichet unique par activité qui s'avérerait complexe à mettre en place notre commission a prévu l'obligation pour l'administration d'orienter, si besoin, le demandeur vers d'autres interlocuteurs administrative dans le mois qui suit sa demande, 20 tiers de cristallisation, l'Assemblée nationale a prévu à l'article 12 bis, une expérimentation que notre commission assorti d'un certain nombre de garanties quant aux 2 autres arguments avancés d'une part, le certificat d'information de l'engagera pas de responsabilités nouvelles de l'administration, puisque comme le site précisément les auteurs, le Conseil d'État a bien rappelé, je cite, qu'en matière de responsabilité de la puissance publique, le projet ne modifie pas l'état du droit, d'autre part je ne saisis pas bien, je suis désolé hein quoi ce certificat sur les compétences d'autres instances, bien qu'est inconsciente délimite dispositif notre commission a donc préféré l'améliorer à l'ouvrage davantage du âgé et en ramenant le délai maximum maximale de réponse à 3 mois plutôt que de le supprimer, vous est donc proposé un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre à vie du gouvernement. C'est un avis défavorable de la même manière, madame la présidente, nous considérons que le certificat d'information est utile pour le lancement de nouvelles activités pour le développement de projets d'entreprise en permettant aux porteurs de projets, disposer d'une information la plus complète possible sur les droits sur la réglementation sur les conditions à observer pour encadrer et accompagner de lancement de cette activité ainsi réduire le risque, ils prennent tout simplement de se tromper, donc l'avis défavorable à la suppression de cet article. Merci, nous allons mettre au voile amendement 142 qui a un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. C'est con. Qui s'abstient l'amendement 142 n'était pas adopté, je mais on voit l'article 12 qui est pour. Qui est con. Qui s'abstient, l'article 12 et d'adopter article 12 bis, nous avons 2 amendements identiques de suppression. Faisant l'objet d'une discussion commune nous commençons par l'amendement 47 présenté par le gouvernement met une mini. En effet, madame la présidente, je rappelé il y a un instant que le certificat d'information a pour objet d'informer les entreprises sur les règles applicables à l'exercice de leur activité, non de se règles comme peut le faire le rescrit la cristallisation pour prendre cette expression du certificat d'information aurait pour effet de permettre aux entreprises de s'affranchir des évolutions juridiques postérieurs à sa délivrance : l'article 12 bis qui fait plus de sécurité pour Biskri pardon : plus mais la cristallisation serait en même temps une source d'insécurité juridique pour les tiers et d'inégalités entre les acteurs économiques intervenant dans un même secteur d'activité, les entreprises exerçant une activité de même nature sur un territoire identiques se verraient appliquer des règles différentes par cristallisation du certificat d'information délivrée et Selosse selon ce selon le moment auquel il aurait été délivrée par ailleurs la cristallisation du certificat d'information pourrait protéger l'entreprise d'une évolution législative quel considérés comme défavorables, de son point de vue, mais pourrait aussi l'empêcher d'avoir accès au bénéfice d'une évolution législative qui seraient favorables favorables au développement de son activité, donc si nous tenons beaucoup au certificat d'information, nous considérons que le cristallisé, comme le propose l'article 12 bis n'est pas opportun, nous en demandons la suppression. Merci monsieur le ministre, nous avons donc la présentation d'une de 2ème amendement identique par monsieur Gontard. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, comme cet article 12 bis est un avatar de l'article 12 que nous avons souhaité supprimer, nous ne pouvons que vous inviter à supprimer également par par cohérence, l'article 12 bis porte sur l'expérimentation d'une forme de durée de validité du STIF certificat d'information document tout de même assez proche d'une fiche de renseignements diffusée en libre accès avec informations sommaires et listes de numéros de téléphone utiles pour renseignements complémentaires qui n'a pas lieu d'être, si l'article n'aient pas introduit dans le droit positif. Monsieur Gontard, avis de la Commission sur ces 2 amendements identiques de suppression. telles qu'introduites sur la proposition du rapporteur à l'Assemblée nationale, je dois avouer que je me suis longuement interrogé au stade de Durban du texte, la commission sur l'opportunité de supprimer une telle expérimentation ou au contraire de la maintenir tout à l'encadrant d'un certaine nombre de garanties, j'ai finalement proposer notre commission qu'il a accepté la seconde option pour les raisons suivantes, qui sont d'ailleurs exposées dans le rapport comme rappelé par le gouvernement dans l'objet de son amendement la cristallisation permet certes de sécuriser juridiquement le détenteur d'un certificat d'information mais comporte, il est vrai, plusieurs risques : le 1er d'entre eux un risque de rupture d'égalité selon qu'on l'aura demandé ou non un certificat d'information, deuxièmement un risque d'effet d'aubaine si d'aventure les usagers les plus avertis multipliait les demandes de certificats dans le seul but de figer les règles, troisièmement, un risque de contournement de normes nouvelles et plus protectrice a matière de santé, de sécurité ou d'un environnement et enfin voir un effet contreproductif consistant à priver le demandeur lui-même de changement de règles qui pourraient lui être favorable, or sur chacun de ces points, il m'a semblé qu'une expérimentation bien encadrés serait malgré tout intéressant d'abord à la tâche à un droit nouveau au certificat d'information, elle lui confère une vraie plus-Value par rapport aux outils de formation existants, ensuite il s'agit bien d'une expérimentation limitée à certaines activités et dans l'évaluation permettra de tirer tous les hein saignement troisièmement la cristallisation des règles existent déjà en matière de certificats d'urbanisme pour une durée du reste plus longue mais celle de a mis ici, sans qu'il ait démontré qu'elle posait problème a en fait un fait notre commission a prévu pour éviter que les dispositions de l'intérêt général puisse être méconnue et s'assurer que la cristallisation sera toujours favorable aux demandeurs, 2 exceptions au profit d'une part des règles préservant directement la santé publique et la sécurité des personnes et des biens ou la environnement et, d'autre part, en cas de demande contraire du détenteur du certificat qui souhaiterait se voir appliquer une règle nouvelle jugée plus favorable, je vous propose donc de maintenir le texte de la Commission et de ne pas adopter ces amendements de suppression d'eau un avis enfin défavorable de la commission. Merci, monsieur le rapporteur, nous avons donc un avis défavorable de la commission ou retrait. Si les 2

Qui s'abstient, l'article 12 bis est adopté article 13 amendements 144 présenté par Monsieur

vous avez la présidente. Alors, la transaction est un mécanisme de règlement des différends relativement peu utilisé par les personnes publiques aurait présente pourtant de nombreux avantages, il ne fait pas obstacle aux peuple et aux prérogatives de l'autorité chargée du contrôle financier ou à une éventuelle saisine du je ne administratif garantissant l'application des règles de droit, or je pense que les dispositions de l'article 13 peuvent réellement favoriser le recours à la transaction et en diminuant aussi les réticences des signataires. C'est pourquoi nous avons cherché à améliorer la rédaction de cet article en commission donc surtout pour que les agents ont fait ne se sentent pas responsables totalement notamment s'ils sont aussi de bonne foi que commettent pas d'erreur, donc je pense que c'est surtout ça qui a amené les agents à ne pas utiliser la transaction, je crois que c'est un moyen aussi important dans ce climat de confiance et et de droit à l'erreur, donc, pour ces raisons-là, nous donnons un avis défavorable à votre amendement Monsieur Bocquet. Merci madame la rapporteur, Monsieur le Ministre à vie du gouvernement. L'avis est défavorable aussi, madame la présidente, dans la mesure où nous partageons les observations faites à l'instant par Madame la rapporteur et un type d'illustrations de souligner qu'en 2016 maisons judiciaire de l'État est intervenu dans 4121 dossiers, au total, seulement 196 ont fait l'objet d'une transaction et notre objectif est bien développé la transaction comme modalité de règlement d'un certain nombre de dossiers, donc l'avis défavorable à la suppression de l'article.

sur le chiffre d'affaires en leur permettant de donner un avis sur les majorations de droits découlant de l'article 1729 du code général des impôts et de la qualification de certaines dépenses de travaux ces commissions sont aujourd'hui au nombre en nombre bien moins élevé qu'auparavant 36 instance au lieu de 101 nous posons donc la question : en quoi l'extension de compétence de ces commissions dont la représentativité et la composition sont tout de même limité apporte un vrai plus aux droits des administrés, nous pensons même certains aspects que cela peut confiner à une forme de mélange des genres qui ne semble pas tout à fait souhaitable un chef d'entreprise désignée par un organisme consulaire pour siéger à la commission pourrait avoir connaissance de la situation d'un de ses concurrents, avec tout ce que cela implique du point de vue de la confidentialité et se pose aussi un problème d'efficacité puisque l'article 1729 s'intéresse singulièrement à la charge de la preuve et à la bonne foi des contribuables puisque les recours gracieux ou contentieux ce fils bien souvent à résoudre les problèmes posés à ce propos, on se rappellera que l'administration traite près de 1,2 1000000 de procédures de recours gracieux et près de 3 millions de procédures en contentieux consistant le plus souvent en un échange d'informations destinée à faciliter la fixation de l'imposition, je ne sais si les commissions ont une activité débordante, eu égard au coût d'ici de saisine, possibilité de récusation ponctuelle, certains mots mais il conviendrait mieux d'assurer, en tous les cas, la présence d'un conseil auprès des contribuables en visite dans les cendres de la DG Philippe de toute autre formule au demeurant réservé ici aux seuls contribuables déclarant des revenus d'activité non salariée et encore ceux qui ont quelques problèmes avec le paiement de leurs impôts, je vous remercie. Merci, cher collègue, avis de la commission Madame Gruny. Merci madame la présidente, alors cet cet article introduit par la commission spéciale et conforme à l'esprit du projet de loi l'application ou non les majorations est il à la bonne foi du contribuable et la qualification d'immobilisation de charges peut relever du droit à l'erreur, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt, sauf à considérer que l'existence même de ces commissions présidées présidées par un magistrat et composé de représentants à la fois de l'administration et des contribuables souvent des Experts comptables souhaitant en elle-même problématique, je crois que sincèrement ces commissions aussi toute leur place en fait pour gérer le contentieux et les les difficultés qui peuvent, qui peuvent être entre les contribuables et l'administration, donc là c'est simplement d'ajouter effectivement le comment le caractère entre immobilisation ou charges déductibles ou alors les majorations de de droit consécutif aux rectifications je pense sincèrement que ça s'intègre bien dans le cadre de de ce texte, donc un avis défavorable à votre amendement moquer. Merci madame la rapporteur, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, après la rapporteure et le rappeler l'article 13 bis étant la compétence des commissions des impôts Directs et taxe sur le chiffre d'affaires qui pourrait désormais se prononcer sur à la fois le caractère d'immobilisation charge une dépense pour l'ensemble des questions relevant de leur Champ de compétences et sur les majorations pour inexactitudes ou omissions dans les déclarations consécutives à des reactif. Question relevant de leur compétence la rédaction qui est adopté par la commission spéciale ne recueille pas véritablement l'assentiment du gouvernement et nous considérons que si le gouvernement doit entendre la demande des sénateurs de travailler sur le rôle de ces commissions, nous devons aussi entendre la demande d'un certain nombre de députés de travailleurs aussi peut-être un peu différemment que ce qui est adopté par la commission spéciale sur le rôle des commissions d'imposition, donc nous souhaitons que la navette parlementaire permette de travailler sur ces différentes hypothèses permettent d'atterrir scolarité sexy cette expression sur un point de consensus à ce stade, parce que nous ne sommes pas convaincu par la rédaction de la Commission, c'est un début de sagesse à l'amendement de suppression proposée par Monsieur le Sénateur bloqué avec cette prévention qui consiste à dire que nous continuons à travailler sur le sujet à l'occasion de la navette parlementaire. Merci monsieur le ministre, je mets aux voix l'amendement 145 qui a donc un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui, pardon

Et Madame, la présidente à Alain, à l'instar de ce qui était prévu à l'article IV en matière fiscale et de contributions indirectes s'agit ici de renforcer la sécurité juridique des contribuables taxes nationales recouvrer, selon les modalités du code des douanes en rendant en rendant t'opposable administration les conclusions, même tacite qu'elle rend à la suite d'un contrôle dans un souci de clarté sur la portée des conclusions de l'administration, il est proposé que les points examinés d'un contrôle, une enquête soit communiquée aux contribuables y compris s'il ne comporte ni erreur ni ni les attitudes ni omission ni insuffisances dans le calcul des droits et taxes éligible cette précision pour nous comme objectif de lever toute ambiguïté sur les points de contrôle entre le contribuable et l'administration des douanes. Il y a avis de la commission madame la rapporteure.

et qui prévoit que les points expressément validé lors d'un contrôle fiscal figurent sur la proposition de rectification, alors ce matin, nous avions demandé le le retrait en raison d'une ambiguïté dans la rédaction, alors après avoir échangé avec le gouvernement, ces difficultés ont été levées, donc je vous propose donc finalement de donner un avis favorable, donc, de ce fait personnelle mais j'engage les membres au moins de la Commission à me suivre. Merci madame la rapporteure, je vais donc mettre aux voile amendement 207 rectifier du gouvernement qui a un avis favorable de la commission qui pour.

dans la droite ligne de l'article de l'amendement pardon qui vient d'être adopté, il s'agit de dire qu'il est prévu lors de la mise en oeuvre la procédure du droit d'être entendu, à la suite d'un contrôle dans douaniers que les conclusions de l'administration porte également sur les points qui l'a examiné, qui ne comporte ni erreur ni ni, ni ni exactitude ni omission ni insuffisances dans le calcul, donc là aussi, c'est pour apporter de la précision et lever toute ambiguïté sur les points de contrôle entre le contribuable e-administration. Merci, monsieur le Ministre, avis de la commission. C'est le même argumentaire, madame la présidente, que pour le précédent, donc c'est un avis aussi favorable. Très bien, merci madame la rapporteure, donc nous mettons voilà Mandement 208 du gouvernement qui a un avis favorable de la commission qui pour.

on va jusqu'à minuit et demi, en fait de demandes de paroles qui sont limitées dans le temps et qui vont se terminer à minuit 30, si vous le voulez, comme ça nous aurons plus qu'à entamer les amendements, demain, je pense qu'on gagne du temps et ça permettra de finir peut-être plus rapidement, si vous en êtes d'accord monsieur nous a, laissons la parole à monsieur courte. Merci madame la présidente, oui je constate pour m'en réjouir qu'effectivement le signal à moitié par le présent article est positif avec l'interdiction pour les administrations d'État, de recourir à un numéro surtaxé, je constate que la rédaction proposée par la Commission va tout à fait dans le bon sens, également, cela fait des années que j'alerte les pouvoirs publics sur la pratique des numéros de téléphone surtaxés plus particulièrement sur ceux à destination des services publics et des services sociaux ou concernant certains organismes transport comme la SNCF dommage d'ailleurs que cet article ne s'applique pas aux établissements publics industriels et commerciaux qu'il me soit permis de faire un bref retour en arrière sur cette question des surtaxés pour rappeler que depuis une dizaine d'années, on les croyait disparus ces numéros surtaxés pourtant depuis peu les voilà subreptice revenu, chacun peut constater en effet que si certaines surtaxes téléphoniques ont baissé ces dernières années en fait dans un grand nombre de cas, la facturation totale de la paix est l'augmentation, la baisse, ce n'était donc illusion en particulier quand l'Otan appelle dépasser les 2 minutes et 20 secondes et faites confiance à certaines de ces organismes, il s'efforce de faire en sorte que l'État n'appel dépasse systématiquement les 2 minutes et 20 secondes Jeanne avait testé quelques heures comme certaines CAF ou à suivre d'assurance maladie ou d'assurance-vie et même encore la SNCF, mieux encore, certains CHU font des économies sur le dos des patients ou de leurs proches, allo service public, c'est la cerise sur le gâteau est un numéro surtaxé, bref de telles pratiques constituent des abus manifestes et pénaliser les personnels de condition modeste, concernant plus particulièrement les services publics, le consommateur paie 2 fois en qualité de contribuable il y a une qualité d'usagers c'est donc aujourd'hui un réel mais pas à n'avoir que nous allons effectuer, avec l'adoption de cet article 15 heures et pour mémoire, nous avons, nous avions effectué un 1er pas avec la loi pour la confiance et dans l'économie numérique, du moins nous le pensions qui prévoyait, dans l'un de ses articles, la gratuité des numéros à destination des services sociaux et il a fallu 7 ans pour que soit publié le décret listant lesdits services sociaux cette année pour faire figurer sur la liste de numéros et seulement 2 numéros désormais gratuit le 115 pour le service d'urgence sans abri et, le 119 pour l'façade nager, alors je ne peux qu'espérer que l'application de l'article 15 heures à sera bien plus rapide, je vous remercie. Oui mais, chers collègues de vous informer que j'avais proposé un amendement à cet article 15 demandant la suppression des numéros surtaxés pour contacter des administrations, cet amendement rapprocher l'entrée en vigueur de cette mesure attendue par nombre de Français de 2021, comme cela est actuellement prévue au 1er janvier 2019, date qui correspond à l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, mesure qui va susciter nombre d'appels qu'elle n'a pas été ma surprise d'apprendre que cet amendement est réputé irrecevables au titre de l'article 40 au motif que cela engendrerait une rupture anticipée des contrats passés entre l'État et les prestataires de services téléphoniques qui ne serait plus honorer et qui donnerait donc lieu à des indemnités, outre le fait que de telles indemnités ne semble pas toujours frappé du recevabilité cet article avait était inséré par voie d'amendements à l'Assemblée nationale avec un gage sans qu'aucune étude d'impact, aucune évaluation disponible du coût de la mesure et des éventuelles indemnités n'été évoqués donc pas débat chiffrées des députés et pas de débat du tout, au Sénat, il aurait pourtant été intéressant de bénéficier de l'évaluation de ses indemnités de rupture pour mesurer la pertinence d'une telle demande et sa mise en oeuvre, tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance, chers collègues, je vous souhaite une bonne nuit. Chers collègues, elle rend maintenant, mesdames et messieurs les sénateurs, je vais lever la séance, nous avons examiné. 60 amendements au cours de la journée, il en reste 112 examiné sur ce texte, ordre du jour du mercredi 14 mars 2018 à 14 heures 30 et le soir, désignation des 27 membres de la mission d'information sur la réinsertion des mineurs ont fermé suite du projet de loi pour un État au service d'une société de. Confiance, la séance est levée, merci à tous.